octobre. Dans la droite ligne du « quoi qu'il en coûte » jupitérien, il n'est quasiment pas une seule journée sans annonce gouvernementale dûment accompagnée d'un chèque à destination d'une partie de nos concitoyens. Chèque énergie, bouclier tarifaire, indemnité inflation : en l'espace de deux mois, vous avez ajouté près de 12 milliards d'euros de dépenses supplémentaires à un déficit public qui s'élève déjà pourtant à plus de 3 000 milliards d'euros, c'est-à-dire 45 000 euros par Français. Je n'ignore pas que ces mesures sont bienvenues dans les foyers français, en particulier chez ceux qui ont l'habitude de gérer leur budget à l'euro près, mais vous n'éteindrez pas leur mécontentement à coups de mesures ponctuelles. Les Français sont lucides, ils ne sont pas dupes, s'agissant, notamment, du poids de cette dette et de la bombe à retardement que celle-ci représente. Alors, monsieur le ministre, face à cette multiplication d'aides ponctuelles, pouvez-vous nous indiquer si le Gouvernement a une stratégie de dépenses publiques ? Plus difficile : quelle sera sa méthode pour assainir les comptes publics ?

Nous avons ensuite proposé à l'Assemblée nationale, qui l'a adopté, un bouclier tarifaire permettant de limiter à 4 % l'augmentation du prix de l'électricité pendant tout l'hiver, mais aussi de plafonner les prix du gaz au tarif du mois d'octobre, afin de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Enfin, face à une inflation plus générale, nous déployons une indemnité inflation de 100 euros pour environ 40 millions de Français, de la manière la plus simple qui soit, puisqu'elle n'aura pas à être demandée et que tout Français gagnant moins de 2 000 euros net par mois en bénéficiera. Ces mesures Ces mesures sont des mesures de protection du pouvoir d'achat et d'accompagnement de la reprise, face à une tension inflationniste liée à cette reprise économique française, européenne et mondiale. Elles sont utiles, et vous avez vous-même rappelé qu'elles étaient bienvenues pour les ménages concernés. Pour ce qui concerne les finances publiques, lorsque nous avons répondu à la crise, nous avons fait le choix du « quoi qu'il en coûte », ce qui s'est traduit par une dégradation du déficit à hauteur de 9,1 % en 2020. Je puis vous assurer, monsieur le sénateur, qu'après toutes les annonces que vous avez rappelées, après toutes les décisions bienvenues pour les Français qu'a annoncées le Président de la République, le déficit public de la France en 2022 sera limité à 5 %. C'est encore beaucoup, certes, mais vous conviendrez avec moi que c'est presque la moitié

de la qualité et de la force de la reprise économique. Nous avons proposé, avec Bruno Le Maire, de revoir le niveau de croissance à 6,25 %. C'est par la croissance, par l'activité, par la richesse produite que nous saurons faire face à cette crise et amortir la dette liée à cette période exceptionnelle. La parole

pas sur le fond, sur les mesures structurelles, sur les renoncements coupables durant les deux derniers quinquennats, du fait de majorités que vous incarnez vous-même parfaitement,

Nous espérons que le Gouvernement ne tardera pas à prendre des décisions pour notre avenir et notre indépendance énergétique, et je sais, madame la ministre, que vous êtes particulièrement sensible à ce sujet. Toutefois, ces scénarios se fondent sur la stratégie nationale bas-carbone, laquelle prévoit une baisse de 40 % des besoins énergétiques français entre aujourd'hui et 2050, ce qui apparaît comme extrêmement ambitieux. RTE mise sur une hypothèse de poursuite de la croissance de 1,3 % à partir de 2030, ce qui se traduirait par une croissance du PIB d'au moins 30 % d'ici à 2050. Dans ces conditions, pour que la consommation d'énergie baisse dans les proportions requises par les scénarios RTE, nous devrions gagner près de 70 % d'efficacité énergétique. C'est colossal, et bien supérieur aux gains observés au cours des trente dernières années. Dès lors, madame la ministre, estimez-vous que cette approche conduisant la France à retrouver son niveau de consommation d'énergie de la fin des années 1960 est plausible ? Comment pourrons-nous concrètement y parvenir ? Quelles décisions, fondées sur les conclusions de ce rapport, avez-vous prévu de prendre ? La parole

Ces travaux confirment qu'il est possible d'atteindre cet objectif tout en maîtrisant la facture des Français ; c'est une excellente nouvelle. Permettez-moi de saluer le travail de concertation très important mené sur deux ans, dont est issu ce rapport. Ce dernier nous indique également quelques constantes importantes. Il est fondé sur une diminution de la consommation d'énergie de 40 % entre aujourd'hui et 2050. Dans le même temps, parce que nous allons décarboner notre mode de vie et sortir de notre dépendance aux fossiles, nous allons électrifier nos usages. La consommation d'électricité va ainsi augmenter de 15 % à 60 % d'ici à 2050, selon les scenarii, en fonction de notre degré de réindustrialisation et de l'évolution des modes de vie. Il faut donc bien distinguer la diminution de la consommation d'énergie en général et l'augmentation de la consommation d'électricité. Votre question porte sur le caractère crédible de cette diminution de 40 % de la consommation d'énergie. C'est cette donnée qui fonde notre stratégie nationale bas-carbone ; elle est ambitieuse, mais elle est dans la ligne des trajectoires européennes et elle peut être atteinte grâce à une efficacité énergétique accrue.

octroyé, depuis le début du quinquennat, 400 000 bonus écologiques et 860 000 primes à la conversion finançant l'achat de véhicules propres et moins consommateurs. Les scenarii de RTE nous donnent donc la possibilité d'atteindre une électricité décarbonée dans une stratégie d'efficience énergétique.

Deuxièmement, nous devons défendre notre modèle au niveau européen, notamment en ce qui concerne la taxonomie. Troisièmement, vous pouvez compter sur le Sénat, en particulier sur sa commission des affaires économiques, pour être une force de proposition pragmatique et sérieuse pour l'avenir de notre indépendance énergétique

Nous adressons toute notre solidarité à sa famille ainsi que nos plus sincères condoléances. Un enfant qui se donne la mort, c'est un drame pour la République et c'est un échec collectif. Nous devons faire en sorte que de tels drames ne se reproduisent pas. Dinah était à un âge où l'on quitte l'enfance, où les projets et les rêves d'avenir se construisent, un âge où la socialisation est fondamentale où, pour ces raisons mêmes, l'on est particulièrement fragile. Il appartient au parquet de Mulhouse d'apporter des réponses quant à la responsabilité de ce drame, mais il semble que Dinah ait été victime de harcèlement scolaire.

Je ne peux parler ici de ce sujet difficile, très délicat, teinté d'une émotion forte, sans évoquer les raisons de ces violences. Celles-ci sont sans doute multiples et complexes, mais je ne peux m'empêcher de m'interroger la banalisation, voire l'acceptation, des discours de haine, d'intolérance et de racisme, particulièrement dans l'arène politico-médiatique, déteint partout, y compris à l'école. Ces problèmes se posent également sur les réseaux sociaux, lesquels, on le sait, ne font guère d'effort pour les modérer. Ce n'est pas une fatalité ; il nous appartient, collectivement, de prendre nos responsabilités. L'éducation de nos enfants, leur émancipation dans de bonnes conditions, est fondamentale ; ils sont notre avenir et l'avenir de notre pays. La parole

elle avait 14 ans. Dans la nuit du 4 au 5 octobre, après deux années d'humiliations quotidiennes, dues à son orientation sexuelle, elle a mis fin à ses jours, comme dix-huit autres victimes de harcèlement scolaire depuis le début de l'année.

Ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est agir avec la plus grande détermination pour que de telles tragédies n'en appellent pas d'autres. Le harcèlement scolaire, véritable fléau de notre société, touche 700 000 élèves, victimes de remarques humiliantes, d'insultes, de menaces, de violences physiques et psychologiques, entraînant des blessures parfois indélébiles. Le cyberharcèlement, lié à la montée en puissance des réseaux sociaux où tout est permis, où, « au fond, rien n'est grave », où l'on oublie l'humain derrière l'écran, accentue ce phénomène.

le harcèlement à l'école et les 10 000 élèves volontaires devenus des ambassadeurs du combat contre le harcèlement. J'en veux enfin pour preuve la directive du 30 septembre dernier visant à mieux accompagner les élèves transgenres, qui a, par ailleurs, fait l'objet de caricatures malheureuses et de polémiques infondées. La lutte contre le harcèlement scolaire, parce qu'elle est intimement liée à notre conception du respect de l'autre, de la réussite éducative, de l'égalité et de l'acceptation des différences, est au coeur de notre projet républicain. Elle passe, bien sûr, par la formation de la communauté éducative dans son ensemble, mais aussi par un partenariat avec les acteurs associatifs, qui se mobilisent chaque jour pour prévenir, pour sensibiliser, pour libérer la parole des enfants, afin de rompre l'insupportable chaîne du silence. Nous le savons, la mobilisation de la société dans son ensemble est essentielle. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelle sera la réponse du Gouvernement afin d'endiguer ce phénomène qui détruit des vies ? La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le

je leur ai demandé de se responsabiliser et de revenir avec des propositions. Nous serons extrêmement exigeants, il y va de l'intérêt de tous. Même les responsables des plateformes le reconnaissent : ils ont, eux aussi, des enfants.

Ces événements tragiques nous révoltent tous. Je vous sais mobilisé sur la question, monsieur le ministre, mais il y a encore des lacunes dans les politiques mises en place. La mission d'information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, que j'ai eu l'honneur de présider aux côtés de la rapporteure Colette Mélot et de tous les groupes politiques de notre assemblée, a unanimement proposé trente-cinq mesures claires et immédiatement applicables. Son rapport a mis en évidence le besoin urgent de renforcement des moyens Les enfants doivent à tout moment pouvoir se livrer à un adulte de confiance, qui donnera suite, et tous les adultes d'un établissement doivent être à même de détecter les signaux faibles. Un renforcement des personnels médico-sociaux, des temps d'échanges dédiés et réguliers, l'utilisation des espaces numériques de travail pour communiquer avec les enfants sur le sujet sont des exemples de dispositifs faciles et rapides à développer.

sur toutes les travées, qu'il est urgent de stopper ce fléau, qui fait encore de trop nombreuses petites victimes. Monsieur le ministre, quand comptez-vous mettre en oeuvre nos propositions ? Quels moyens d'envergure entendez-vous déployer pour réagir, et réagir vite ?

à de très nombreuses reprises ces derniers temps. Nous allons étoffer les équipes d'intervention extérieure des rectorats vers les établissements, lorsque ces phénomènes se produisent, et les établissements sont évalués, dès maintenant, sur l'enjeu du climat scolaire. je voudrais dire que la question de l'engagement des adolescents, notamment à partir du collège, dans des causes d'intérêt général fait aussi partie de la solution, parce que nous devons développer des logiques de fraternité et de non-violence dans nos établissements. Cela passe aussi par les aspects positifs de l'engagement de nos élèves. La parole

la présomption forte d'un lien entre l'exposition professionnelle aux pesticides et six pathologies graves. On connaît aussi l'impact des perturbateurs endocriniens. La question cruciale est donc celle de l'après. Que ferons-nous de ces chiffres, qui vont jeter l'opprobre uniquement sur les agriculteurs ? Demain, comment l'Anses, qui est juge et partie, car elle autorise la mise sur le marché de ces produits, va-t-elle diffuser des éléments à charge ? ma question est double : cette étude est-elle lancée uniquement en France ou également dans d'autres pays européens viticoles ? Comment allez-vous anticiper l'annonce de ces résultats, qui vont, une fois encore, placer les paysans au banc des accusés, alors même que ceux-ci ne font qu'utiliser des produits homologués et autorisés, et alors que la filière viticole s'inscrit depuis des années dans des démarches durables avec différents labels,

elle est arrivée dans sa phase de déploiement et va durer trois ans ; ses résultats sont donc attendus pour 2024. Comme toute étude scientifique, celle-ci se doit d'être objective, neutre et rigoureuse.

bio dans notre pays a doublé depuis 2017. Nous sommes devenus le pays européen avec la plus grande surface biologique. Le label HVE est très utilisé dans le domaine viticole. Le nombre d'exploitations qui s'y soumettent a été multiplié par

continuent à dire que l'agroécologie ne serait pas une réalité sur le terrain ! Monsieur le sénateur, soyez certain que la science doit être là pour éclairer, pour progresser et jamais pour caricaturer. Telle devra être

sur les réseaux sociaux, qui sont eux aussi aux mains de quelques milliardaires et dont les algorithmes sont incontrôlables, ainsi que le révèlent les. Dans ce

qu'avez-vous fait pour respecter l'engagement pris par Emmanuel Macron en 2017 de protéger l'indépendance éditoriale des médias ? Qu'avez-vous fait pour lutter contre la concentration des médias, préservant ainsi une condition essentielle pour la démocratie et un débat public apaisé ?

Outre la concurrence exacerbée qui règne habituellement, l'apparition des grandes plateformes numériques et des réseaux sociaux y participe Nous avons besoin de champions nationaux forts pour pouvoir investir massivement dans la création, à la fois française et européenne. doivent toutefois se dérouler dans le respect du pluralisme et de la diversité de l'offre, qui sont d'ailleurs des principes garantis par la Constitution.

il nous faut bien constater- nous partageons ce diagnostic -que les textes qui assurent cette régulation sont déjà anciens

à réduire de moitié les usages des produits phytosanitaires et, surtout, à diminuer de 10 % les surfaces cultivées sur notre continent. De nombreuses études, dont celle du Centre commun de recherche de la Commission européenne, mettent en avant les effets potentiellement négatifs de cette stratégie. La Commission a malheureusement maintenu sa ligne directrice initiale, sans mener d'étude d'impact sérieuse. On estime les pertes de production entre 15 % et 20 %, ce qui aura des conséquences sur le revenu des agriculteurs. De plus, devrait faire face à une situation de dépendance alimentaire. D'exportateurs, nous pourrions devenir importateurs net. Toujours selon la même étude, l'impact sur la lutte contre le changement climatique serait très faible. il s'agit là, bien évidemment, de l'objectif recherché ! Monsieur le ministre, ces propositions font fi de la situation géopolitique et sont à contre-courant des ambitions que nous portons pour l'agriculture européenne. Ce renoncement stratégique

Ne faisons pas à notre agriculture ce que nous avons fait à certains pans de notre industrie ! Très bien ! L'agriculture doit poursuivre sa transition progressive, sans brutalité, en mobilisant la recherche et l'innovation. Monsieur le ministre, vous aurez dans quelques semaines la lourde responsabilité de présider le conseil des ministres de l'agriculture de l'Union européenne. Quelle ligne défendrez-vous pour garantir durablement la souveraineté alimentaire de l'Europe ?

La nouvelle politique agricole commune va tellement loin que, comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, la production diminuera

Alexandra Borchio Fontimp, pour le groupe Les Républicains.

Nous sommes le 27 octobre, la saison a démarré, comme vous le savez, et les professionnels ne connaissent toujours pas les conditions d'accès aux remontées mécaniques, alors que vous vous étiez engagé à leur apporter des réponses claires avant la mi-octobre. Les maires des stations de montagne, les dirigeants des remontées mécaniques sont désabusés. Ils ont à présent besoin de savoir de manière extrêmement claire quel sera leur mode de fonctionnement. Élue des Alpes-Maritimes, je compte dans mon département sept stations de ski, dont certaines se remettent à peine de la tempête Alex.

on reste évidemment bien plus éloigné des autres que sur une plage, dans un centre commercial ou dans une rame de métro. Les acteurs du tourisme hivernal comptent sur cette saison pour rebondir. Ils sont las de vos atermoiements et de votre manque d'anticipation et de lisibilité- ce sont décidément les éléments caractéristiques de votre gestion de crise. préférez-vous, une fois de plus, annoncer vos décisions aux directeurs des remontées mécaniques, quelques heures avant leur mise en application ? Monsieur le ministre, pouvez-vous définitivement nous rassurer, cet après-midi, dans l'hémicycle, quant à l'avenir de nos stations de ski ?

et Républicain. Ma question s'adresse à Mme la ministre déléguée chargée de l'industrie. Le 15 octobre dernier, le groupe finlandais UPM a annoncé son choix de céder le site de Chapelle Darblay, à Grand-Couronne, en Seine-Maritime. L'avenir de ce site n'est pas une affaire locale. L'usine est la dernière en France à être en capacité de produire du papier 100 % recyclé. Elle dispose d'une puissance de recyclage de 480 000 tonnes par an, soit la collecte effectuée auprès de 24 millions de Français, dans un périmètre de 400 kilomètres incluant l'Île-de-France. Le projet retenu par UPM, celui du groupement Samfi-Paprec, comprend une activité de tri des déchets sans recyclage, l'utilisation d'une chaudière biomasse et l'hypothétique mise en place, d'ici trois à cinq ans, d'une unité de production d'hydrogène. Une offre alternative, portée par Veolia et Fibre Excellence, a été écartée. Pourtant, celle-ci prévoit la production de 400 000 tonnes de cartons d'emballage, dont la demande explose, à partir des papiers et cartons usagés, collectés en France. Elle permet la préservation du site industriel, des machines, des compétences et recrée 250 emplois. Elle utilise la voie fluviale et constitue un projet cohérent d'économie circulaire. Elle a le soutien des syndicats, qui ont fait preuve de responsabilité dans ce dossier, et des élus locaux. La métropole Rouen Normandie entend faire valoir son droit de préemption. Madame la ministre, il faut préserver l'outil industriel et éviter le démantèlement des machines. Comment le Gouvernement compte-t-il intervenir et appuyer la démarche de la collectivité ?

Cette boussole, je le sais, est aussi celle des élus du territoire, des représentants du personnel et des anciens salariés. Grâce à notre mobilisation,

Marie, pour la réplique. Madame la ministre, depuis l'arrêt des machines, 480 000 tonnes de papier ont été envoyées à l'étranger, incinérées ou enfouies. Dans sa présentation du plan France 2030, le Président de la République a insisté sur la nécessité d'investir dans le recyclage et il a fait de l'économie circulaire une priorité. L'initiative de la métropole Rouen Normandie doit donc être appuyée par le Gouvernement. Des instructions doivent être données pour éviter le démantèlement du site. Des discussions doivent être de nouveau engagées avec UPM pour que l'offre alternative soit sérieusement examinée. La réindustrialisation du pays et le développement de l'économie circulaire nécessitent que le Gouvernement passe des paroles aux actes. La parole est à M. Hugues Saury, pour le groupe Les Républicains. l'économie, des finances et de la relance. Le démarchage téléphonique peut être un véritable fléau et confiner au harcèlement. C'est la raison pour laquelle le système concessif nommé « Bloctel » a été mis en service en 2016. Plus de 4 millions de foyers y ont recours, pour environ 11 millions de numéros de téléphone.

Depuis quatre ans, et contractuellement jusqu'à mai 2021, la société Opposetel avait la charge de ce service. Avec plus de cinq mois de retard, la société Wordline a finalement été désignée pour une durée de cinq années.

Ensuite, il semblerait que les consommateurs inscrits sur cette liste constatent une recrudescence d'appels intempestifs. Enfin, les entreprises qui adhèrent au dispositif et paient un abonnement ne parviennent plus, quant à elles, à identifier les numéros qui leur sont interdits et risquent, dès lors, de se voir infliger une sanction pouvant aller jusqu'à 75 000 euros

Cette mobilisation s'applique en particulier à la lutte contre les sollicitations téléphoniques indésirables. Le démarchage téléphonique non sollicité est un désagrément majeur pour nos concitoyens, parfois dérangés plusieurs fois par jour. Je suis, comme vous, pleinement conscient de l'attente extrêmement forte des Français dans ce domaine. Pour améliorer le service tant pour les consommateurs que pour les entreprises, un nouveau prestataire a été récemment retenu à l'issue d'un appel d'offres. Mis en place depuis le 1 octobre ce nouveau prestataire modernise le service pour proposer davantage de fonctionnalités à un coût nettement plus limité pour les entreprises, en particulier les plus petites. Ce changement de prestataire et les travaux de modernisation en cours ont une incidence logique, mais temporaire sur le service, même si tout est fait pour qu'elle reste la plus limitée possible. Dès le début de l'opération, les consommateurs inscrits sur Bloctel ont continué d'être couverts par le service, puisque leurs numéros avaient été retirés des listes de démarchage traitées au mois de septembre.

Depuis le 25 octobre, il est de nouveau possible de s'inscrire pour protéger son numéro. Les services de la DGCCRF sont en contact régulier avec les associations de consommateurs et les entreprises du secteur pour les tenir informées en toute transparence de l'avancée des travaux. Monsieur le sénateur, je peux vous assurer que les services de la DGCCRF sont totalement mobilisés pour faire, par ailleurs, cesser le démarchage abusif.

appels d'offres qui ont été lancés par l'État. Le premier concernait la distribution des tracts électoraux, le second porte sur Bloctel. Vous avancez des arguments pour expliquer ces dysfonctionnements, mais, une fois encore, le constat reste que le défaut de pilotage politique, associé à la lourdeur administrative,

Une nouvelle fois, le rapport est accablant. Sur 129 produits testés, 60 % présentent une anomalie et 32 % sont même dangereux. La totalité des dispositifs médicaux testés présentaient un défaut. Serions-nous impuissants à protéger nos concitoyens ? La DGCCRF indique qu'elle a immédiatement fait retirer les produits concernés de la vente en ligne. C'est une goutte d'eau dans un océan d'impunité Sur 15 adaptateurs électriques, 13 présentent un danger de choc électrique pour le consommateur. Combien de produits, qui sont aujourd'hui vendus en ligne, présentent un risque, en particulier pour les enfants ? Le problème est aussi économique, car une concurrence déloyale s'installe entre les charlatans qui oeuvrent et les commerçants de nos territoires qui paient des loyers, des charges sociales, des taxes foncières et qui respectent les normes. Les commerces, touchés durant la crise sanitaire, ne peuvent pas continuer d'être concurrencés par des plateformes qui menacent la sécurité des consommateurs et qui profitent de l'ampleur des flux pour inonder notre pays de produits dangereux et non conformes. Monsieur le ministre, face au constat que la DGCCRF a établi depuis plus de deux ans, quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour que les produits vendus sur internet respectent les mêmes normes que ceux que l'on trouve dans les magasins ? Comment ferez-vous pour imposer des sanctions dissuasives ?

Il s'agit, par exemple, de bijoux fantaisie qui contiennent trop de métaux lourds, de chargeurs de téléphone susceptibles de déclencher des incendies, ou encore de peluches mettant en danger la vie des enfants. Les places de marché en ligne sont une formidable opportunité pour de nombreuses PME, notamment françaises. Le revers de la médaille est qu'en développant ce modèle économique on facilite l'accès à notre marché national de vendeurs implantés dans des pays tiers, qui ne sont pas toujours au fait des règles européennes de protection des consommateurs.

le Président de la République. La DGCCRF exerce une vigilance constante pour suivre l'état du marché et faire retirer les produits dangereux. Monsieur le sénateur, soyez assuré de la totale détermination du Gouvernement, en particulier de Bruno Le Maire et Cédric O, pour avancer vite et fort sur cette question.

pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, le Gouvernement a lancé, le 19 octobre dernier, les Assises de la forêt et du bois, sous l'égide de quatre ministères. La biodiversité devient un enjeu primordial et la décarbonation, un principe directeur des orientations budgétaires. craignons néanmoins que la lutte contre les incendies n'ait été oubliée. Pourtant, les conséquences des méga-feux sont considérables. L'incendie du Var a ravagé 7 000 hectares en quatre jours, produisant 325 000 tonnes de CO2, l'équivalent de six mois d'émissions dans les transports de l'agglomération marseillaise.

Alors que la guerre du feu requiert des moyens aériens en adéquation avec la recrudescence des incendies sur le pourtour méditerranéen, notre flotte de Canadair est vieillissante. Son renouvellement est possible dans le cadre d'une commande collective permettant la réouverture des chaînes de production. L'Europe pourrait se doter alors d'une flotte d'appui aux pays méditerranéens, avant que l'inéluctable changement climatique n'affecte aussi des territoires plus septentrionaux. Dans le cadre de la troisième convention des maires de la région Sud, j'ai fait part au président de la commission du développement régional du Parlement européen de cette nécessité de constituer une force d'intervention européenne. fort de ces constats, je souhaite vous poser deux questions. Le Gouvernement est-il prêt à intégrer la problématique du feu dans le cadre des Assises de la forêt et du bois, et à soutenir les collectivités dans la mise en oeuvre des actions de prévention ? ? La présidence française de l'Union européenne peut-elle permettre d'engager la mise en place d'une flotte aérienne européenne de bombardiers d'eau, qui complétera et renforcera la nôtre ?

que la moitié d'entre eux sont dus à des imprudences. Il faut sans cesse le dire et alerter sur ce point. Avec le ministre de l'intérieur, nous renforçons également les moyens de détection, en développant des systèmes plus efficaces pour faire remonter sans délai les premiers signaux de départs de feu et limiter la propagation. Avec le ministre de l'agriculture, nous travaillons à rendre plus effectives les obligations légales de débroussaillement.

et Républicain. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il s'écrit actuellement en Nouvelle-Calédonie un chapitre politique majeur. À la suite de l'accord de Nouméa, signé par Lionel Jospin dix ans après les accords de Matignon conclus par Michel Rocard- vos prédécesseurs -, deux référendums se sont tenus et ont montré l'attachement de la Nouvelle-Calédonie à la République française. Le troisième référendum est prévu le 12 décembre prochain. Nous savons tous que ce scrutin se tiendra dans un contexte international et régional tendu. Considérons d'abord le contexte international. Nous assistons depuis plusieurs années à la multiplication d'opérations de déstabilisation électorale de grande ampleur référendum sur l'indépendance de l'Écosse en 2014, présidentielle états-unienne de 2016, alertes récentes d'une ancienne employée de Facebook, pour ne citer que ces trois exemples. Ces attaques contre le libre arbitre des citoyens sont des maux mondiaux, que l'on ne peut ignorer, surtout dans le climat de tension que connaît la zone indo-pacifique. J'en viens ainsi au contexte régional. L'Indo-Pacifique est en proie à de très fortes tensions. Les prises de position américaines récentes contre la puissance chinoise et les retournements d'alliances dont la France a fait les frais placent ce scrutin référendaire dans un environnement que l'on ne peut ignorer. Ne doutons pas que l'ensemble des puissances régionales s'y intéressent de très près. Nous souhaiterions donc connaître, monsieur le Premier ministre, votre appréciation s'agissant des risques d'ingérence étrangère dans cette campagne référendaire. que vous nous précisiez les moyens mis en oeuvre pour y faire face. Enfin, pouvez-vous nous indiquer les mesures prises par votre gouvernement pour assurer un bon déroulement du vote, afin de garantir une légitimité irréprochable à ce scrutin ?

Depuis quelques semaines, ceux-ci interpellent de nouveau, manifestent, proposent, cherchent en vain à être entendus. Ils sont effectivement sûrs d'une chose : ils ne pourront refaire une saison comme celle qu'ils viennent de vivre, avec des attaques de loups incessantes sur des territoires de plus en plus étendus. Cette année, au-delà des habituelles brebis et chèvres, ce sont déjà une centaine de vaches et de veaux qui ont été victimes du prédateur dans mon seul département, ainsi que des chevaux, ânes et chiens. Que dire quand des agriculteurs n'ont pas d'autre choix que d'achever eux-mêmes le travail du loup sur des animaux qu'ils ont élevés avec soin ? Est-ce du bien-être animal ? Est-ce du bien-être au travail ? ? L'entêtement de Mme la ministre à gaspiller de l'argent public- les indemnisations coûtent de plus en plus cher -, à être dans ce contresens écologique est incompréhensible. Protection, « quoi qu'il en coûte », d'une espèce ; disparition de combien d'autres ? Il n'y a plus un seul mouflon en Haute Maurienne depuis que les loups s'y sont installés. On peut aussi parler de la flore surpiétinée dans les enclos de nuit loi Climat et résilience qui favorise le consommer local et durable, ce que nous appelons de nos voeux, et il empêche en même temps nos éleveurs de produire laitages et viandes. Leurs demandes sont simples : un comptage contradictoire, la responsabilité en justice de l'État pour les chiens qui leur sont imposés

qui doivent prévoir des mesures au plus près, de l'effarouchement aux prélèvements éventuels. Ces mesures doivent effectivement constituer des réponses adaptées, rapides et territorialisées. Nous y travaillons. Parce que le comportement des prédateurs, la topographie des territoires ou encore le type d'élevages

tout à fait présent aux côtés des agriculteurs et des éleveurs pour l'indemnisation des pertes liées à ces attaques. C'est un impératif, mais ce n'est évidemment pas suffisant. Nous avons donc demandé,

Le préfet coordonnateur a rassemblé autour de lui tous les préfets dédiés ... Il faut conclure ! ... pour maintenir ce pastoralisme dans nos territoires, tout en respectant et en assurant la préservation d'une espèce essentielle aux équilibres des écosystèmes.

l'ensemble de notre biodiversité, et non pas une seule espèce, qui compte plus à vos yeux que la détresse de nos éleveurs et de leurs familles. La

Une page de la presse locale de mon département m'a interpellée. Elle rapporte que l'insuffisance cardiaque est la première cause d'hospitalisation après 65 ans. Ce mal insidieux, qui touche un Français sur cinq, doit être dépisté le plus tôt possible pour éviter une aggravation de la maladie. Si l'insuffisance cardiaque n'est pas traitée, elle entraîne la mort dans 50 % des cas. On estime que 1 % à 2 % de la population française est concernée, soit 1,4 million de personnes. À titre de comparaison, c'est autant que la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, on meurt moins du cancer du sein que d'une insuffisance cardiaque. Nous savons que cette maladie touche plus les femmes que les hommes. Les hospitalisations pour insuffisance cardiaque aiguë sont au nombre de 160 000 et on peut comptabiliser 70 000 décès à l'échelle d'une année. Pourtant, le grand public ignore encore largement cette affection. Il y a urgence à organiser un dépistage précoce de la maladie et à créer une filière de soins spécifiques. Nous devons absolument en connaître les signes sans les banaliser. Il est de notre devoir de communiquer au grand public cette information. Madame la ministre, cela est-il une priorité de santé publique ? Si oui, tous les hôpitaux sont-ils dotés d'un service de cardiologie ?

en médecine de premier recours. Ainsi, nous avons inscrit le repérage du risque cardiovasculaire dans les politiques de formation continue des soignants, afin que les médecins sachent mieux accompagner les personnes à risque. À titre d'exemple, nous valorisons également un projet expérimental de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, l'AP-HP, qui permet une meilleure coordination des intervenants à l'usage de la télésurveillance, l'optimisation thérapeutique par transfert de compétences, etc. Je citerai aussi le projet As qui permet le développement de l'activité physique adaptée pour les patients insuffisants cardiaques et qui est développé dans de nombreux territoires. Nous souhaitons enfin lancer très prochainement une mission sur les mobilités actives,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

indélébile dans le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour consolider les acquis, pour réparer les injustices, pour réduire les inégalités, chaque mesure et chaque voix comptent. effet, au pays de l'égalité, il est insupportable que les femmes, qui représentent la moitié de l'humanité, restent victimes de discriminations, de violences et de préjugés qui les empêchent de s'accomplir. En tant que responsables politiques, nous avons donc l'impérieuse responsabilité de faire de l'égalité- en l'occurrence, de l'égalité économique et professionnelle -une réalité concrète et effective. Alors qu'un vent de conservatisme s'est levé sur l'Europe et sur le monde, mettant en péril les droits des femmes, pourtant conquis de haute lutte- un vent qui ne s'arrête pas aux frontières de l'Hexagone -, nous devons au contraire accélérer. Avancer plus vite sur le chemin de l'égalité constitue justement l'antidote face à la montée des radicalités et des relativismes, car il est des combats qui rehaussent une nation tout entière, des combats qui doivent tenir lieu d'horizon : le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes est de ceux-là. Avant d'aborder plus en détail le texte qui nous réunit, permettez-moi de rappeler quelques chiffres. À poste équivalent et à compétences égales, l'écart salarial entre les femmes et les hommes atteint 9 % dans notre pays. Pas moins de 78 % des emplois à temps partiel, qui sont majoritairement subis, sont occupés par des femmes. les femmes ne représentent que 30 % des dirigeants d'entreprises et à peine 12 % des créateurs de start-up dans le secteur d'avenir qu'est la. la. Elles touchent des retraites inférieures de 42 % en moyenne à celles que perçoivent les hommes. Ces inégalités ne sont plus acceptables, alors que les femmes ont été et sont encore en première ligne face à la triple crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons. Rétablir l'égalité, ce n'est donc pas leur accorder une faveur. Rétablir l'égalité, ce n'est pas leur accorder la charité. Rétablir l'égalité, c'est réparer une injustice que rien ne saurait justifier, une injustice hier tolérée, mais devenue aujourd'hui

les moins reconnus et les moins valorisés ! Non, les femmes ne doivent pas accepter d'être absentes de la table où se prennent les décisions ! Aujourd'hui, il n'y a plus ni excuse ni prétexte. Oui, nous avons besoin de tous les talents pour redresser notre économie. Oui, nous avons besoin que les femmes soient présentes dans les filières scientifiques et dans les métiers d'avenir des nouvelles technologies. Et oui, face aux inégalités et aux discriminations, c'est toute cette assemblée et toute notre société qui doivent faire bloc ! Car l'égalité ne se décrète pas. Elle ne jaillit pas d'un claquement de doigts dans une société qui demeure, à maints égards, patriarcale et sexiste. Elle se construit et sexiste. Elle se construit pas à pas, notamment grâce à la loi. La proposition de loi qui nous réunit ce soir embrasse un large spectre de l'égalité économique entre les femmes et les hommes. De l'aide aux familles monoparentales jusqu'à la place des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, en passant par l'entrepreneuriat féminin et la création de viviers de talents dans l'enseignement supérieur, ce texte s'adresse à toutes les femmes de notre pays et à toutes les générations.

Alors que les femmes sont aussi formées, compétentes et ambitieuses que les hommes, comment expliquer cette disparité si importante ?

C'est pourquoi je suis favorable aux mesures contraignantes visant à accélérer l'accession des femmes aux postes stratégiques dans les entreprises. Les quotas ne sont antinomiques ni avec la méritocratie ni avec la reconnaissance des compétences et des talents. Ils sont au contraire des accélérateurs de cette méritocratie. La loi du 27 janvier 2011, dite « loi Copé-Zimmermann », dont nous avons fêté les dix ans cette année, est l'illustration concrète que les quotas fonctionnent. Grâce à elle, la France est devenue championne d'Europe en matière de féminisation des conseils d'administration de ses grandes entreprises. Il s'agit là d'une fierté collective, collective, qui fait rayonner notre pays au-delà de ses frontières. Mais nous devons aujourd'hui aller plus loin pour transformer durablement notre société et la rendre enfin plus inclusive. Nous devons parallèlement continuer à mettre en oeuvre des dispositifs permettant de traiter à la racine les mécanismes qui reproduisent les inégalités. C'est l'objet de plusieurs autres articles de cette proposition de loi ; je m'en réjouis. loi ; je m'en réjouis. Au cours de ma vie antérieure en entreprise, j'ai pu constater que l'un des obstacles majeurs à la progression des carrières des parents est l'accès à une solution de garde pour les enfants. C'est un fait établi, en particulier pour les familles monoparentales, qui sont à 85 % composées d'une femme avec enfants : rappelons que 700 000 d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Sur l'initiative d'Adrien Taquet, le Gouvernement a réduit le coût des assistantes maternelles, notamment pour les femmes seules avec enfants, en augmentant de 30 % le montant du complément de mode de garde. avec les collectivités territoriales, le soutien à la création de nouvelles places de crèches dans les quartiers défavorisés. proposition de loi soutient clairement les familles monoparentales en leur réservant des places en crèche afin de leur permettre de trouver un emploi, de créer une activité, ou encore de participer aux actions d'accompagnement professionnel.

mais il est indispensable que celles qui le souhaitent ne soient pas bloquées par des préjugés sexistes et que leur liberté d'entreprendre ne soit pas entravée par des stéréotypes de genre d'un autre temps.

j'ai récemment renouvelé avec Bpifrance l'accord-cadre relatif à la promotion et au financement de l'entrepreneuriat féminin dans les territoires. En effet, il est crucial

Comme vous le voyez, les acteurs publics sont donc extrêmement engagés sur ce sujet. Mesdames, messieurs les sénateurs et sénatrices, le temps de l'égalité concrète et effective est venu. Les nouvelles générations nous le demandent.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il y a dix ans, nos prédécesseurs votaient la loi Copé-Zimmermann.

de la proposition de loi de la députée Marie-Pierre Rixain, de franchir une nouvelle étape en permettant aux femmes de prendre toute leur place

m'ont dit qu'ils avaient hâte que les femmes prennent toute leur place dans les instances dirigeantes des entreprises, qu'ils jugent eux-mêmes trop masculines. J'aborde donc ce texte avec la conviction que l'égalité

venir au détail de ce texte, son premier volet vise à favoriser l'égalité salariale. Depuis 2019, les entreprises doivent publier un index de l'égalité professionnelle, qui comporte cinq indicateurs. Celles qui n'atteignent pas un score doivent prendre des mesures correctrices ; une pénalité financière est prévue au bout de trois ans. Cet index est à nos yeux un levier efficace en faveur d'une meilleure égalité salariale, même s'il est encore trop tôt pour en évaluer pleinement les effets. C'est pourquoi la commission considère

Les entreprises qui n'atteignent pas le score global de 75 sur 100 devront également définir et rendre publics des objectifs de progression pour chaque indicateur. J'en viens au deuxième volet du texte, à savoir le partage des postes à responsabilité. La loi Copé-Zimmermann n'a pas eu d'effet sur les postes décisionnels à l'intérieur de l'entreprise. Concrètement, les femmes représentent 46 % des membres des conseils d'administration des grandes entreprises, mais

dans le texte que sur les quotas fixés et le calendrier retenu. Je vous proposerai donc de conserver cet équilibre. Concernant la publication des écarts de rémunération sur le site du ministère du travail, la commission propose qu'elle soit effective dans cinq ans, c'est-à-dire au moment de l'entrée en vigueur des premiers quotas.

proposition de loi, Bpifrance devra en outre rechercher un équilibre hommes-femmes parmi les bénéficiaires de ses actions, d'une part, et au sein de ses comités d'investissement, d'autre part. La commission a énoncé plus clairement l'objectif chiffré de 30 % de femmes au sein des comités d'investissement, tout en fixant l'échéance de 2025 pour y parvenir. Enfin, les financements de Bpifrance seront conditionnés à la publication, par les

Au-delà de ces sujets liés à l'entreprise, la proposition de loi concerne aussi d'autres aspects de l'égalité professionnelle : l'autonomie financière des femmes, la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, ainsi que l'égalité des chances dans le système éducatif. d'autonomie financière, la commission a apporté des précisions aux articles 1 et 2, qui prévoient l'obligation de verser le salaire, ainsi qu'une liste de prestations sociales, sur un compte bancaire dont le salarié ou le bénéficiaire Elle a également adopté l'article 1 , qui permet l'exercice du « droit au compte » afin de permettre à des femmes victimes de violences de s'extraire de l'emprise financière de leur conjoint.

pour les femmes enceintes. Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait un droit à douze semaines de télétravail avant le début du congé maternité. Il nous a semblé que cela risquait d'éloigner

La commission propose que ce sujet fasse partie des négociations sociales et soit intégré dans les accords sociaux d'entreprise ou dans les chartes sur le télétravail. Le texte aborde aussi l'égalité des chances dans l'enseignement supérieur, en se fondant sur l'idée que c'est en amont de l'entreprise qu'il faut former un vivier de femmes susceptibles d'accéder à tous les métiers. La commission a approuvé l'article 5, qui oblige les établissements de l'enseignement supérieur à publier des indicateurs sur l'égalité entre hommes et femmes pour chacune de leurs formations. Elle a également approuvé les mesures visant à renforcer la parité des jurys de concours et de sélection, ainsi que la publication d'indicateurs sur l'égalité au sein des établissements de recherche. Enfin, la commission a supprimé du texte les précisions sur la lutte contre les stéréotypes de genre dans l'enseignement secondaire et dans ses liens avec l'enseignement supérieur, considérant que toutes ces dispositions étaient déjà satisfaites par le droit en vigueur. En conclusion, mes chers collègues, il apparaît que cette proposition de loi comporte plusieurs outils pour améliorer la place des femmes dans l'entreprise et dans la société. Le Président Jacques Chirac avait l'habitude de dire que le degré de civilisation d'une société se mesure à la place qu'y occupent les femmes. Cette jolie phrase signifie non seulement que la place laissée aux femmes reflète la qualité d'une vie en société, mais aussi- et c'est ma conviction ! -qu'elle y contribue fortement. La commission vous propose donc d'adopter ce texte, en formant le voeu qu'il fasse avancer notre société tout entière. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je me réjouis que notre assemblée examine aujourd'hui cette proposition de loi déposée par mon homologue, Mme Marie-Pierre Rixain, présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, qui est présente dans nos tribunes Nos deux délégations ont travaillé parallèlement, en bonne intelligence, sur le sujet important de l'accès des femmes aux responsabilités au sein des entreprises. Je tiens à remercier sincèrement notre rapporteure Laurence Garnier, qui a été à l'écoute des préoccupations de notre délégation et avec qui nous avons pu échanger afin d'améliorer encore cette proposition de loi. Il s'agit d'un texte majeur. Dix ans après la loi Copé-Zimmermann, qui a introduit des quotas de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance, il est en effet nécessaire de franchir une étape supplémentaire.

montré que les quotas ont fonctionné, mais qu'ils n'ont pas eu l'effet de ruissellement attendu. Alors que les femmes représentent 46 % des membres de conseils d'administration et de surveillance des entreprises du SBF 120- les 120 plus grosses entreprises cotées françaises

La parité est encore plus limitée dans les instances de gouvernance et de direction des entreprises à petite capitalisation boursière et des entreprises non cotées. Forte de ces constats, notre délégation avait formulé des recommandations afin d'étendre les obligations de parité et de mixité et de renforcer le contrôle du respect des obligations existantes. Nous soutenons donc pleinement les dispositions de la proposition de loi en la matière, en particulier son article 7, qui introduit des quotas de femmes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des entreprises de plus de 1 000 salariés. nous souhaiterions que le calendrier retenu soit accéléré. Il faut cesser de repousser les échéances. La loi Copé-Zimmermann a prouvé que le vivier de femmes compétentes était bien là.

De même, le baromètre Sista sur les conditions d'accès au financement des femmes dirigeantes de start-up indique que les équipes masculines représentent 85 % des start-up financées et 90 % des fonds levés en 2020.

Enfin, j'aimerais dresser quelques perspectives pour les années à venir. Je pense qu'il nous faudra nous pencher à nouveau sur l'index de l'égalité professionnelle. C'est un excellent outil qui a permis à de nombreuses entreprises de prendre conscience de certains dysfonctionnements. Ainsi, 13 % des entreprises n'appliquent pas encore l'augmentation de salaire au retour de congé maternité qui est pourtant prévue par la loi depuis 2006. Nous sommes convenus qu'il est encore trop tôt pour modifier les indicateurs au sein de cet index, que toutes les entreprises doivent s'approprier, mais il faudra y réfléchir. Je pense notamment à un indicateur permettant de mettre en lumière la surreprésentation des femmes parmi les 10 % des rémunérations les plus basses, ou encore à un autre sur le nombre de pères qui utilisent pleinement leur congé paternité, dont je souhaiterais d'ailleurs allonger la durée, notamment pour ce qui est des jours obligatoires. En effet, c'est dès les premiers jours de l'enfant que se répartit la charge parentale. En En attendant ces discussions futures, je me réjouis d'entamer l'examen de cette proposition de loi. Le Sénat s'honorera de voter ce texte, qui marque une étape importante pour la progression de la place des femmes et des responsabilités qui leur reviennent au sein de nos entreprises. Il faut enfin faire exploser le plafond de verre de la direction opérationnelle des entreprises ! Bravo ! Avant de

Monge. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j'aimerais tout d'abord saluer le travail de la commission des affaires sociales et celui de Laurence Garnier, rapporteure de cette proposition de loi qui vise à accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Je veux également saluer l'action de la délégation aux droits des femmes du Sénat, qui alimente abondamment nos réflexions sur ces sujets si importants.

Son périmètre est par nature limité ; pourtant, elle touche un sujet qui aurait mérité qu'on s'y attarde longuement : comment bâtir une économie qui prenne en compte les différences entre les femmes et les hommes ? Il existe en effet une différenciation fondamentale, la maternité, laquelle impacte forcément, de manière concrète, la vie des femmes. Abolir cette différence n'a pas de sens ; il faut l'accepter et réfléchir en profondeur pour bâtir une économie soucieuse de cette différence : je pense en particulier à l'impact du congé

l'instauration de quotas a donné des résultats et a permis sa féminisation. Je suis pour la méritocratie : ne devrait-on pas choisir un employé selon ses compétences personnelles, selon ses mérites, plutôt que selon son sexe ou son origine ethnique ? Aucune femme n'a envie d'être nommée à un poste uniquement parce qu'elle est une femme : la compétence opérationnelle doit primer. Nous ne pouvons douter des progrès réalisés en matière d'égalité.

depuis la mise en oeuvre de ce texte. Ainsi, la France se situe au premier rang mondial en termes de féminisation des conseils d'administration des grandes entreprises, avec une proportion de 46 % de femmes en 2021. La délégation a aussi souligné que la parité restait limitée dans les conseils d'administration des plus petites capitalisations boursières et, plus globalement, des PME. Il n'y a donc pas eu de ruissellement des instances de gouvernance vers les instances dirigeantes des entreprises, ce qui plaide pour une extension de la logique des quotas. J'ajoute que, à poste équivalent, les femmes gagnent en moyenne 10 % de moins que les hommes. Ces inégalités ne sont pas acceptables. Améliorer la place des femmes dans la société et dans les entreprises en favorisant leur progression et notamment leur accès à des postes à hautes responsabilités est donc une nécessité. En outre, l'égalité femmes-hommes est une source de performances et de succès pour nos entreprises. Cette proposition de loi permet donc d'avancer ; j'en partage bien évidemment les intentions générales. J'attire cependant l'attention sur le fait que les formalités obligatoires supplémentaires qu'elle crée pour nos entreprises ces dernières, en tout cas certaines d'entre elles qui font d'ailleurs un certain nombre d'efforts pour maîtriser le fonctionnement de l'index Egapro introduit récemment, en 2018. Certaines entreprises sont aussi préoccupées par le cumul des sanctions. Il est important de trouver des solutions équilibrées, mais notre rapporteure a oeuvré en ce sens. Traiter de l'égalité par le biais de quotas est donc une réponse partielle à un problème complexe qui trouve ses origines dans la culture, dans l'orientation à l'école, dans la formation, dans la gestion des talents et dans l'évolution des carrières. Je pense aussi à la nécessité de renforcer la mixité dans les sciences, les technologies et l'ingénierie, domaines où l'on sait qu'il y a pénurie de femmes alors que les besoins de recrutement sont extrêmement importants.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dix ans après la loi Copé-Zimmermann, le temps était venu d'une évaluation et d'une loi ambitieuse pour un beau combat celui de l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce texte n'y suffira pas, mais il comporte des avancées. Selon l'Insee, le revenu salarial net des femmes représente 71 % de celui des hommes et les mêmes inégalités se retrouvent, très aggravées, pour les retraites et le patrimoine. Dans les entreprises, la présence des femmes diminue au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie et les inégalités salariales se creusent au long du parcours professionnel. Si la France se situe aujourd'hui à la première place en Europe en matière de féminisation des conseils d'administration des grandes entreprises cotées, dépassant même le quota obligatoire, l'effet d'entraînement attendu au niveau des instances de direction des entreprises, lieux des décisions stratégiques et opérationnelles non couverts par ces obligations,

Les articles relatifs à l'index de l'égalité professionnelle- extension de son champ, publicité des indicateurs, des mesures de correction et des objectifs de progression -vont dans le bon sens, mais cet outil n'est vraiment qu'une première étape que, faute de nouvelles perspectives, des entreprises risquent de considérer comme une fin en soi. en soi. Pourtant, des scores suffisants au regard des exigences légales peuvent masquer la persistance d'inégalités non questionnées, notamment dans le champ de la formation continue et des promotions, inégalités dues en partie aux biais et aux stéréotypes de genre. Cela entretient la faible mixité de certains postes, fonctions et emplois, facteur d'inégalités structurelles dont ne rend pas compte le seul principe « à travail égal, salaire égal »- ce principe n'est d'ailleurs pas respecté, de la mesure de priorisation des places en crèche pour les familles monoparentales- de fait, des femmes -, nous y sommes favorables. Mais il faut bien dire que nous gérons seulement la pénurie alors que manquent des solutions de garde pour tous les enfants. Cela appellerait la mise en place d'un service public de la petite enfance, enfance, levier majeur pour l'égalité. Concernant l'obligation de verser les salaires et les prestations individuelles sur des comptes dont la personne est titulaire ou cotitulaire, nous demanderons, au nom du principe de précaution, de ne pas interdire la désignation d'un tiers par mandat écrit. l'autonomie financière doit aussi être pensée avec et pour les femmes en situation de pauvreté ou de grande pauvreté. Évitons qu'une mesure positive ne devienne un obstacle de plus dans leur quotidien quand le droit à un compte bancaire est encore loin d'être effectif dans notre pays. Ces mesures sont précieuses dans la lutte contre la violence économique au sein des couples ; rappelons combien le refus du Gouvernement d'individualiser l'allocation aux adultes Alors que, le temps d'une crise sanitaire, la situation des femmes a reculé et qu'ont été effacés les progrès réalisés depuis plusieurs années en France- et depuis plusieurs décennies dans le monde -, nous refusons

En effet, seul ce niveau de discussion permet d'aborder toutes les situations, notamment celles des femmes occupant des postes ne pouvant être exercés en télétravail, qui sont souvent les plus pénibles, et de s'assurer des conditions du volontariat.

chers collègues, que l'égalité professionnelle est inscrite dans la loi du 13 juillet 1983, la loi Roudy ? Depuis lors, de nombreuses lois ont été votées pour garantir l'égalité des droits, dans l'entreprise, entre les femmes et les hommes. Et pourtant, rien n'a changé, ou si peu, pour la plupart d'entre elles. La loi Copé-Zimmermann de 2011 a imposé aux entreprises de plus de 500 salariés une représentation de 40 % de femmes dans les conseils d'administration, alors qu'elles comptaient jusqu'alors pour moins de 10 %. Dix ans après, on estime à 44,6 % la proportion d'administratrices dans les grandes entreprises. Certes, c'est un progrès indéniable, mais ces chiffres masquent mal la réalité du quotidien de la grande majorité des femmes de notre pays. Ainsi, l'égalité économique et professionnelle visée par la proposition de loi ne concerne qu'une minorité de femmes, celles qui exercent leur activité dans les grandes entreprises. Or 67 % des femmes travaillent dans les secteurs de l'administration publique, de l'enseignement, de la santé et de l'action sociale. Je rappelle que 97 % des aides à domicile sont des femmes, de loi de financement de la sécurité sociale prévoit l'instauration d'un tarif plancher à 22 euros, mais c'est largement insuffisant pour augmenter le salaire de ces femmes et cela ne résout pas la question de l'amplitude horaire très large et morcelée de leur travail pour des salaires de misère.

Ce texte fait totalement l'impasse sur la précarité du travail féminin, la sous-valorisation de ces métiers, ou encore l'absence de formation pour des centaines de milliers de femmes, pourtant en première ligne contre la pandémie de covid-19, qui vivent avec moins de 700 euros par mois. Vous allez me dire que ce n'est pas l'objet de cette proposition de loi ; mais alors, pourquoi lui avoir donné un tel titre ? Les mots ont un sens ! Une fois encore, ces femmes sont les grandes oubliées, les invisibles de la société. Une proposition de loi qui ne cible qu'une minorité de femmes, cadres dans des entreprises de l'assurance ou de la finance, semble bien éloignée, madame la ministre, du moment historique pour l'égalité entre les femmes et les hommes D'autant que, selon un rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) d'avril dernier, en un an de crise sanitaire, on a perdu près de trente ans d'avancées dans le domaine de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi, en 2021, les femmes subissent encore des rémunérations inférieures aux hommes- à poste et qualification égaux -pouvant aller jusqu'à 24 %. Les femmes demeurent davantage touchées que les hommes par la précarité, le temps partiel et le chômage, leurs carrières sont davantage plafonnées, elles accèdent moins souvent aux postes de responsabilités. Elles sont également plus discriminées en raison de leur genre et s'occupent davantage que les hommes des tâches domestiques et de l'éducation des enfants.

si la création d'un index de l'égalité est une bonne mesure, force est de constater que sa conception même en fait presque un gadget. L'égalité professionnelle et économique va bien au-delà de cet index ; il y a urgence à adopter des mesures pour lutter contre la précarité et le temps partiel, à créer une place d'accueil pour tous les enfants de moins de trois ans et à revaloriser les métiers à prédominance féminine. Hier, la délégation aux droits des femmes du Sénat récompensait par un prix un certain nombre de personnalités ayant fait progresser les droits des femmes.

Alors que les femmes représentent 33,72 % des cadres de ces mêmes entreprises, 22,37 % seulement sont membres de leur comité exécutif. Cette proposition de loi, à défaut de grands progrès, apporte de petites améliorations pour renforcer la parité dans l'exercice du pouvoir. Je regrette que la rapporteure Laurence Garnier l'ait affaiblie en supprimant un certain nombre de dispositions introduites par l'Assemblée nationale. De même, je regrette que la question de l'impact des violences domestiques sur les salariés n'ait pas été considérée comme entrant dans le périmètre de cette proposition de loi. Bref, le chemin vers l'égalité semble encore loin

de débattre d'une proposition de loi sur l'égalité économique et professionnelle ? J'aurais pu d'ailleurs utiliser un autre terme, mais je m'en suis privé ... Ma réponse est « oui », doublement « oui » : l'égalité entre les femmes et les hommes est un fait de société qui nous concerne toutes et tous, même si je dois confesser que, pour moi, cette question relève plus de la conversion que de la conviction spontanée- je suis plutôt saint Paul que saint Pierre en la matière ... C'est sans doute pour cette raison que, dans une volonté de travailler sur moi-même, j'ai récemment lu plusieurs ouvrages sur ce sujet. Je voudrais en citer un aujourd'hui, à savoir le livre passionnant de Frédéric Dabi,, qui traite de l'évolution de de l'opinion des jeunes depuis les années 1960. Parmi les chiffres marquants qui ont retenu mon attention, il y a celui-ci : 72 %- oui, 72 % ! -des 18-30 ans estiment qu'il est plus facile d'être un homme qu'une femme.

parce que c'est un problème qui me paraît facile à résoudre. Et là, maintenant que je suis grande, je me rends compte que ce problème n'est toujours pas réglé. » Oups ! Alors, bien sûr, c'est simplement dit et la réalité est souvent plus complexe. Mais cela ne change pas le problème de fond. Dans ce même livre, Frédéric Dabi confirme un sentiment personnel que j'éprouve depuis longtemps : les jeunes ne sont pas dans la logique du « tous pourris » ou dans une logique générationnelle, comme on peut l'entendre ici et là ; ils sont plutôt dans une logique de défiance par rapport à l'impuissance publique. Ils veulent des résultats et j'ai pour espoir qu'avec ce texte, même si beaucoup de choses restent à faire, nous pourrons commencer à apporter des résultats en la matière. Je souhaite saluer l'esprit du présent texte ; la loi Copé-Zimmermann a plus de dix ans aujourd'hui et il est essentiel de proposer une nouvelle loi en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je suis heureux aussi que, sur ces questions, nous puissions trouver un consensus entre les différents groupes de notre assemblée, car l'égalité entre les sexes est un enjeu majeur. Aujourd'hui, cela devient même, me semble-t-il, un enjeu de civilisation et notre capacité à résoudre ces injustices sera déterminante dans le regard que porteront les futures générations sur notre action.

l'entrepreneuriat féminin. J'ai été particulièrement marqué par un chiffre mentionné dans l'excellent rapport de notre collègue Laurence Garnier : 80 % des fonds investis dans les start-up françaises ont été dirigés vers des équipes intégralement masculines en 2020. Ce chiffre donne à réfléchir : sommes-nous incapables, en France, d'investir dans nos talents féminins ou, pis encore, sommes-nous incapables de donner aux jeunes femmes de notre pays l'envie de s'engager dans une aventure aventure entrepreneuriale ? L'égalité entre les hommes et les femmes ne s'inscrit pas uniquement dans le respect des droits ou dans les postes de cadres en entreprise, mais aussi dans le lancement de projets,

aux banques privées et aux fonds d'investissement. La seconde disposition que je souhaite saluer est celle qui entend favoriser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, notamment en ce qui concerne la garde d'enfants et la parentalité. C'est entre trente et quarante ans que se forge une carrière, mais aussi que les femmes

C'est en train de changer », dit-elle, ajoutant que « les entreprises sont conscientes qu'il faut changer les règles du jeu ». Elle conclut : « Je suis optimiste pour l'avenir. » Je partage cet optimisme et j'espère que nous y contribuerons par cette proposition

disposition qui m'interpelle : la diffusion par le ministère du travail des scores obtenus par les grandes entreprises, selon la pratique dite du « ». Personnellement, je vous le dis, mes chers collègues, je ne soutiens pas ce type de pratique. Bien sûr, je peux en comprendre l'utilité et la capacité d'influence, mais il ne me semble pas que ce soit le rôle de l'État

à accompagner la parentalité et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Il n'est donc pas nécessaire d'inscrire dans la loi les dispositions proposées alors que ces associations diffusent déjà une information sur ces stéréotypes.

je vous remercie

chers collègues, si du temps a passé depuis la loi Copé-Zimmermann- dix ans, pour être précise -, le constat reste le même : à travail égal et à ancienneté égale, une femme reste toujours moins bien payée qu'un homme.

Ensuite, il y a une répartition des métiers qui fait que les femmes font le choix de carrières souvent moins bien rémunérées que celles des hommes. Enfin, il y a une part qui reste non identifiée, qui est celle de la discrimination à proprement parler, parfois inconsciente, mais bien réelle pour les femmes qui la subissent. S'il y a eu de récentes évolutions- je pense notamment à l'allongement du congé paternité -, certains freins persistent, notamment en matière de responsabilités. C'est vrai aussi C'est vrai aussi bien en entreprise qu'en politique : si la parité au sein des assemblées délibérantes et des exécutifs est actée, seulement 11 % des présidents d'exécutif sont des femmes. Pour en venir à cette proposition de loi, si le travail de la commission est venu clarifier le texte sur certains points, celui-ci n'apporte pas de révolution majeure : nous sommes loin de la grande cause du quinquennat ! Au titre des déceptions, on note surtout la consécration de droits non opposables, comme cela a déjà été dit. Je pense notamment à l'article 4 sur l'accès des familles monoparentales aux modes de garde collectifs, qui ne crée pas d'obligation, malgré le manque de places dans de nombreuses villes. Ce n'est pas un service public, me direz-vous, mais au vu de l'ampleur des places manquantes, il faudra un jour s'interroger sur la manière dont les pouvoirs publics peuvent investir ce sujet. Au titre des dispositions ne créant pas d'obligations, nous avions une véritable interrogation sur les douze semaines de télétravail pour les femmes enceintes, prévues initialement à l'article 3 . Si le dispositif pouvait être intéressant pour les femmes concernées, il comportait plusieurs risques : d'abord, celui qu'il soit très fortement proposé- pour ne pas dire imposé -à une femme et qu'il vienne remplacer le congé maternité. Ensuite, il créait une inégalité mesure où toutes les femmes ne disposent pas d'emploi leur permettant de télétravailler. Concernant l'article 1 relatif au versement des salaires et des prestations sociales de manière individualisée, nous y sommes favorables, mais nous regrettons que la majorité de l'Assemblée nationale se contredise, à en juger par son vote sur la déconjugalisation de l'AAH. Finalement, les Finalement, les véritables avancées proposées à ce texte se trouvent à l'article 7, qui prévoit d'étendre l'objectif de représentation équilibrée aux instances dirigeantes d'une entreprise. Nommer et blâmer les entreprises qui ne respecteraient pas cet impératif de 30 %, puis de 40 %, de femmes dans les instances dirigeantes est, selon nous, une nécessité. Pendant trop longtemps, nous en sommes restés à l'incitation ; il est désormais nécessaire d'agir plus intensément pour faire bouger les lignes : c'est ce qui nous est proposé à cet article 7. Nous proposerons aussi, par voie d'amendement, de rétablir la version de l'Assemblée nationale pour que la publication des éventuels écarts se fasse un an après l'entrée en vigueur de cette loi et non pas cinq ans après, comme le propose la commission. À cet article 7, toujours, nous proposerons également d'instaurer un plancher pour le montant des pénalités prévues en cas de non-respect des obligations de représentation de chaque sexe au sein des postes à fortes responsabilités. Pour conclure, le groupe du RDSE, dans sa majorité, votera ce texte, conscient qu'il n'apporte pas de grandes révolutions, mais estimant qu'il représente un pas supplémentaire dans la longue marche vers l'égalité entre femmes et hommes en entreprise. La parole

l'engagement, la détermination et la sincérité de Mme la ministre et vous dire, madame, le plaisir que nous avons- que j'ai, en tout cas -à travailler avec vous et à défendre ensemble, de concert, la cause des femmes. Vous aurez compris, à cet instant, que je vais dire

Le Gouvernement avait en effet promis à plusieurs reprises de faire progresser l'émancipation économique des femmes ; finalement, dans ce texte, les ambitions de la majorité s'articulent autour de quelques ajustements, de quelques renforcements des dispositions d'égalité professionnelle et d'une grande mesure- disons-le - : l'instauration des quotas dans les comités exécutifs, mesure que je ne sous-estime pas et dont je ne néglige pas la portée aujourd'hui et, surtout, à l'avenir, non pas simplement pour les femmes membres de ces comités, mais aussi pour son effet « montant » dans les entreprises et la nécessité pour les dirigeants de chercher des viviers pour répondre à ces futures obligations. Cependant, alors que les plans de relance consécutifs à la crise sanitaire auraient pu être les vecteurs d'un déploiement massif de financements facilitant l'égalité entre les femmes et les hommes- ce que nous proposions d'ailleurs avec le collectif Ensemble contre le sexisme dans l'« appel des 40 pour un plan de déconfinement antisexiste

Cet état de fait, dont tout le monde admet l'injustice, doit cesser. S'il était bon que la loi de 1972 sur l'égalité des salaires en affirme le principe, il manquait à cette loi les moyens réels d'application des principes qu'elle pose. » Cette phrase est extraite du discours prononcé par Yvette Roudy, en 1982, pour présenter la loi sur l'égalité salariale.

Nous avons progressé à petits pas. Les écarts de salaire ont diminué, mais ils restent très importants, de l'ordre de 20 %. Les femmes sont toujours moins bien payées que les hommes ; elles sont plus souvent à temps partiel, par choix ou non, d'ailleurs ; elles sont davantage exposées à la précarité, ce qui rend plus difficile la défense de leurs intérêts collectifs.

Ces inégalités se sont fortement accentuées avec le confinement. Les difficultés spécifiques des femmes pendant la crise sanitaire ont déjà été évoquées. Toutefois, rappelons que les femmes sont majoritaires dans de nombreux métiers clefs,

43 % des salariées françaises envisagent un temps partiel, contre 32 % des hommes. Les femmes constituent aussi la majorité des personnes en situation de précarité. Les statistiques sont implacables

il faut que le monde professionnel cesse de faire des économies sur le dos des femmes. Il est plus que temps, dirai-je même, de leur rendre l'argent ! L'égalité économique et professionnelle des femmes et des hommes est un droit. Chaque avancée législative, chaque nomination de dirigeantes au sein des instances de gouvernance des entreprises, chaque condamnation pour discrimination à l'embauche en raison du sexe, chaque mesure de rattrapage salarial est une petite victoire de plus glanée au service d'un idéal, celui de l'égalité. En créant un quota dans les comités exécutifs, le présent texte poursuit le chemin ouvert par les lois précédentes. Nous y sommes favorables. Les élus du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ont par ailleurs déposé un certain nombre d'amendements visant à améliorer cette de renforcer les obligations paritaires des entreprises ou de faciliter l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Toutefois, nous regrettons certaines modifications opérées en commission, qui atténuent fortement la portée du texte. Les mesures de lutte contre les stéréotypes sexistes dans l'enseignement secondaire et supérieur sont amoindries. Pourtant, c'est lors de l'orientation que s'enclenchent bien des mécanismes qui privent plus tard les filles de l'accès aux domaines d'activité les plus rémunérateurs, aux emplois techniques et aux fonctions de pouvoir. La publication de l'ensemble des indicateurs de l'index égalité pour le secteur privé est de surcroît repoussée

aucune disposition n'est prévue pour le public. Or la fonction publique attend toujours des améliorations, alors que l'État employeur devrait être exemplaire. Les résultats obtenus en matière de féminisation de l'accès aux emplois d'encadrement supérieur et dirigeant s'améliorent, mais ils restent trop contrastés. quel que soit le volontarisme politique de cette proposition de loi, puis de son application, l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes ne sera pas atteint tant que les violences sexuelles et sexistes infligées aux femmes ne seront pas éradiquées. À ce titre, je regrette l'absence de dispositions de protection des femmes face aux violences, alors même que le monde professionnel pourrait

ce texte aurait pu être l'occasion de créer de nouveaux congés pour événements familiaux, une dispense de préavis pour démission ou encore une protection contre le licenciement. Ce sont là des solutions pragmatiques, utiles immédiatement pour des victimes qui doivent déjà suivre un parcours difficile, mais salutaire, vers la sortie des violences. Mes chers

il y a dix ans, la loi Copé-Zimmermann imposait des quotas de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance des grandes entreprises. À l'époque, il s'agissait de franchir une étape décisive dans le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette législation faisait de la France un pays avant-gardiste en la matière.

s'agisse des revenus- à poste égal, les femmes gagnent 10 % de moins que les hommes et seules 6 % des entreprises françaises versent des salaires égaux -, de la sécurité au travail- 30 % des Françaises ont déjà été harcelées ou agressées sexuellement sur leur lieu de travail-, de la formation- en 2018, les femmes ne représentaient que 34 % des bénéficiaires de contrats d'apprentissage dans le secteur privé -, du financement- elles ont 30 % de chances en moins d'être financées par les principaux fonds de capital-risque que les hommes

Face à ce constat, le Gouvernement a pris des engagements forts en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans un certain nombre de secteurs. Je pense à la fonction publique, avec la loi du 6 août 2019, qui favorise l'égalité professionnelle et la prévention des discriminations, notamment en instaurant un plan pluriannuel visant à garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique. Je pense à l'enseignement supérieur et la recherche, avec la loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020. Je pense également au monde de l'entreprise, avec la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a créé l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce dernier exemple illustre la nécessité d'aller encore plus loin. En effet, si 70 % des entreprises ont publié leur index en 2021, seulement 56 % des entreprises affichent un score supérieur à 75.

Je pense, enfin, à l'allongement du congé de paternité, véritable outil au service de la justice sociale : cette mesure permet d'assurer un rééquilibrage des tâches familiales et, partant, de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, même si, à titre personnel, je souhaiterais que nous allions plus loin C'est dans ce contexte que nous examinons la proposition de loi de notre collègue Marie-Pierre Rixain, laquelle permet de franchir une étape supplémentaire, dans la continuité des réformes engagées. Son adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale envoie un message fort à la société,

Il améliore le droit au compte, même en cas de compte joint, pour assurer aux salariées une maîtrise de leurs revenus. Cette garantie est essentielle, notamment en cas de violences conjugales : grâce à elle, les femmes ne seront plus dépendantes financièrement de leur conjoint violent.

Il améliore également la transparence de l'index de l'égalité professionnelle et permet un meilleur accès des femmes aux fonds d'investissement. Ce faisant, il tire les conséquences de la situation actuelle. il vise à renforcer la parité dans les instances dirigeantes, dans la continuité de la loi Copé-Zimmermann. Je tiens à saluer le travail de la rapporteure et l'esprit qui a guidé nos votes en commission afin de préserver l'équilibre du texte. y a apporté un certain nombre de modifications. Je pense par exemple à l'article 8, qui introduit des objectifs de mixité dans la politique de soutien à la création et au développement d'entreprises et précise l'entrée en vigueur de certaines dispositions prévues.

Il s'agissait d'une réelle avancée, au regard des effets positifs du télétravail sur la néonatalité, à la fois pour la santé des mères et pour les nouveau-nés.

Le présent texte est issu de cet engagement. Il vient compléter les mesures prises par le Gouvernement à la suite du Grenelle contre les violences conjugales, comme le bracelet anti-rapprochement, par des dispositions visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les hommes et les femmes. Le constat est sans appel : à poste équivalent, les femmes gagnent en moyenne 10 % de moins que les hommes. La raison principale est le recours au temps partiel. Les emplois dont il s'agit sont occupés à 80 % par des femmes, dans une société où la répartition des rôles au sein de la famille reste inégalitaire et marquée par des stéréotypes tenaces. Il est de la plus grande importance de faciliter autant que possible la conciliation entre l'activité professionnelle et la vie familiale des femmes, en particulier pour les familles monoparentales, tout en renforçant la féminisation des postes à responsabilités et de certaines filières pour atteindre une représentation plus équilibrée des femmes dans la société. des travaux de l'Assemblée nationale contient d'importantes avancées favorisant l'émancipation financière et professionnelle des femmes. Il s'attaque au plafond de verre, qui ferme un certain nombre de postes à responsabilités aux femmes, en instaurant un objectif clair : atteindre, en 2030, 40 % de femmes parmi les cadres dirigeants des entreprises de plus de 1 000 salariés. La loi Copé-Zimmermann a imposé cet objectif pour les conseils d'administration des entreprises et, avec dix années de recul, nous savons que ce dispositif fonctionne. un autre plan, l'épreuve de la crise sanitaire a démontré, en généralisant le télétravail à grande échelle, qu'une autre forme d'organisation du travail était possible. Nous savons que de nombreux salariés ont apprécié les effets positifs du télétravail sur leur qualité de vie. Il a notamment limité les temps de transport et la fatigabilité associée. Ce qui est vrai pour de nombreux salariés l'est davantage encore pour les femmes enceintes et pour les jeunes parents. laquelle je souhaite rétablir l'article 3 , adopté par l'Assemblée nationale, mais supprimé par notre commission des affaires sociales. Cet article instaurait un droit au télétravail pour les femmes enceintes douze semaines avant leur congé de maternité. je vous proposerai d'aller plus loin, en étendant cette possibilité après l'accouchement, seize semaines suivant la fin du congé de maternité. Avec ces amendements, je vous proposerai d'adopter une mesure concrète qui bénéficiera à de nombreuses femmes dont les missions peuvent être effectuées à distance. En créant un droit au télétravail, nous améliorons la qualité de vie des femmes enceintes et nous facilitons le recours à l'allaitement pour les femmes qui le souhaitent.

l'employeur serait en droit de refuser une demande de télétravail si les fonctions occupées par la salariée ne pouvaient pas être exercées à distance. Ces dispositions très concrètes seraient sans conséquence sur les finances publiques ou sur les finances de l'entreprise. En revanche, elles représenteraient une avancée considérable considérable en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comme en matière de santé publique. « Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les franchir ; vous n'avez qu'à le vouloir dès 1791, Olympe de Gouges, première des féministes, plaçait l'émancipation des femmes au coeur de notre

les femmes sont une catégorie à part et ce qu'il faut arriver à faire justement, c'est qu'elles cessent de l'être ». Prononcée par Françoise Giroud, première secrétaire d'État à la condition féminine, en 1974, cette phrase est encore criante de vérité et d'actualité. La proposition de loi examinée aujourd'hui par notre chambre vise à accélérer l'égalité professionnelle et économique entre les femmes et les hommes : c'est une grande ambition et un honorable objectif que de parvenir, par exemple, à un équilibre parfait dans la représentation des femmes au sein des instances dirigeantes.

Ainsi, je ne peux que saluer les avancées notables de ce texte pour lutter contre les violences économiques faites aux femmes, les accompagner lorsqu'elles sont engagées dans un parcours d'insertion professionnelle, instaurer des mécanismes de comptage des hommes et des femmes et, enfin, combattre les stéréotypes de sexe, notamment dans les établissements d'enseignement supérieur.

Toutefois, le constat est sans appel : les femmes demeurent exclues des fonctions à hautes responsabilités. On le voit clairement : l'accès des femmes à ces postes ne se fait pas au fil du temps par autorégulation des acteurs. Elle ne peut advenir qu'en étant imposée par des quotas assortis de sanctions. On le vérifie dans de nombreux cas, en particulier dans la sphère politique là où la loi sur la parité ne s'applique pas, les femmes sont sous-représentées. Dès lors, continuons à faire évoluer nos lois pour enfin permettre une véritable représentativité de la société Si les quotas sont efficaces pour atteindre la parité numérique, ils ne sont pas l'unique solution pour l'égalité. Ils n'en constituent pas moins un outil indéniable au service du progrès social. Instaurer des quotas ne revient pas à privilégier une femme au détriment d'un homme, mais au profit d'une assemblée, d'un territoire ou d'une entreprise. Les femmes sont plus diplômées, mais moins représentées, surtout lorsqu'il s'agit de postes à grandes responsabilités :

et toujours, cette situation en 2021, c'est continuer à donner des gages à la discrimination. Or l'égalité, comme la liberté, ne s'accorde pas à moitié, elle doit être pleine et entière. On n'est pas à moitié égal ou à moitié libre : puisque l'organisation spontanée ne parvient pas à garantir l'égalité pleine et entière, la seule réelle, c'est le rôle de la loi de corriger ce mécanisme discriminatoire. Les quotas sont le seul moyen démocratique d'y parvenir, car ils produisent un effet immédiat d'égalité. C'est une pierre supplémentaire que nous nous apprêtons à poser en votant ce texte : de telles dispositions sont nécessaires à l'édifice que nous bâtissons et il est certain que nous continuerons ce combat, femmes et hommes, ensemble ! Très bien

cet enjeu majeur transcende les différents pans de notre société. De nombreuses évolutions, notamment législatives, ont déjà permis des avancées considérables, mais nous savons que le combat de l'égalité demeure un combat permanent d'une part, rien n'est jamais acquis dans ce domaine ; d'autre part, il est indispensable d'accompagner les avancées nouvelles. La proposition de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, que nous examinons aujourd'hui, est un nouveau pas à saluer, et j'en remercie son auteur, le députée Marie-Pierre Rixain. Je tiens également à souligner le travail de notre collègue rapporteur, Laurence Garnier, qui a contribué, grâce à de nombreuses auditions, à donner une portée réelle et concrète d'être une femme reste le premier facteur d'inégalité dans l'environnement professionnel. Cette inégalité prend souvent racine dès la formation et l'orientation, avant de perdurer tout au long de la carrière.

Dans le même temps, il ressort d'un récent rapport de la délégation sénatoriale aux droits des femmes que la loi de 2011 n'a pas entraîné une féminisation de la gouvernance et de la direction de toutes les entreprises. Le constat est clair : la parité reste limitée dans les conseils d'administration des plus petites entreprises non cotées de plus de 250 salariés. Les femmes accèdent moins souvent que les hommes aux comités les plus stratégiques et les plus rémunérateurs. Le plafond de verre

texte impose une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les cadres dirigeants des entreprises. En ce sens, il répond à la fois à une réalité et à un besoin. Je salue son caractère réaliste, ambitieux

ma part, j'insisterai sur deux points qui me paraissent particulièrement importants. Le premier, c'est le rôle clef de l'orientation. Le choix des études et d'une profession reste très sexué ; ainsi, 50 % des femmes se concentrent sur 15 % des métiers.

En renforçant l'égalité des chances dans le système éducatif et dans l'enseignement supérieur, ce texte va dans le bon sens. D'ailleurs, de nombreuses initiatives locales existent en la matière, à l'instar du prix régional

paraît donc plus appropriée. Mes chers collègues, nous avons un devoir collectif : tout faire pour parvenir à une égalité réelle en donnant les mêmes chances et les mêmes possibilités aux femmes et aux hommes. C'est ce à quoi nous invite cette proposition de loi en matière professionnelle et économique.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement du groupe Écologiste- Solidarité et Territoires vise à permettre au salarié de désigner, par mandat écrit uniquement, un tiers pour recevoir son salaire.

étant, l'interdiction de désigner un tel tiers pourrait porter préjudice aux personnes en situation de pauvreté ou de grande pauvreté. Les associations

du Gouvernement ? Vous l'aurez compris, madame la sénatrice, l'objectif de cet article est de protéger les femmes qui sont déjà victimes de violences. Même si j'entends les arguments que vous nous opposez, je suivrai Mme la rapporteure en émettant un avis défavorable.

montre bien le lien entre travail, déplacements et prématurité.

Il s'agit d'améliorer les conditions de travail des femmes enceintes et de favoriser la poursuite du travail jusqu'au moment du congé de maternité, un mois et demi avant le terme. le terme. Ce nouveau droit me semble tout à fait justifié ; il correspond aux évolutions actuelles de la société en matière d'organisation du travail et d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des femmes. Nous souhaitons rendre pleinement effectif le droit à l'allaitement inscrit dans le code du travail, à raison d'une heure par jour répartie entre le matin et le soir, en ouvrant un droit au télétravail jusqu'à six mois après la naissance. Il ne s'agit pas de confondre télétravail et garde d'enfant, car les femmes auraient bien entendu la possibilité de faire garder leur enfant à domicile pendant les horaires de travail, comme cela est de plus en plus pratiqué avec le développement du télétravail. Les femmes sont actuellement confrontées à un choix difficile entre poursuite de l'allaitement et reprise du travail, ce qui incite les jeunes mères soit à renoncer à l'allaitement exclusif les six premiers mois, soit à retarder la reprise de leur activité professionnelle. La société évolue, tout comme les modes d'organisation du travail : il nous semble que notre rôle est d'accompagner ces changements. Cette disposition aurait un impact positif à trois égards elle renforcerait l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en favorisant la conciliation entre travail et maternité ; elle améliorerait le niveau de santé publique puisque, je le rappelle, l'allaitement maternel est un facteur protecteur contre un certain nombre de maladies pour l'enfant et la mère ; enfin, elle constituerait une mesure de politique familiale favorisant la maternité sans pénaliser le travail. est à Mme Guylène Pantel. Cet amendement tend à accorder aux femmes enceintes qui le demandent un droit au télétravail dans les douze semaines précédant le congé maternité, lorsque cela est possible. Plusieurs études, dont une menée au Danemark et une autre en Irlande, ont en effet montré que le recours au télétravail imposé par la pandémie avait eu un effet positif sur la santé des futures mères et des futurs nouveau-nés. Le confinement a conduit à une diminution du nombre de naissances prématurées. Les chiffres restent certes approximatifs, puisque certains hôpitaux français ont estimé cette baisse à 20 % et d'autres à 15 %. Il semblerait toutefois que le télétravail permette aux futures mères de travailler dans un cadre moins bruyant et moins stressant, et de limiter les trajets qu'elles doivent sinon accomplir pour se rendre sur leur lieu de travail. Le télétravail favoriserait ainsi des grossesses plus saines et moins éprouvantes. Les

3 concernant les femmes enceintes. L'objectif initial de la disposition introduite par l'Assemblée nationale était de permettre aux femmes enceintes de bénéficier d'un droit au télétravail douze semaines avant leur congé maternité. Le bénéfice de cette forme d'organisation du travail est évident pour la santé de la salariée

Nous avons vu que le télétravail lié au confinement a surgi dans les entreprises, contribuant à un nouveau mode de travail. S'il a pu présenter un certain nombre d'opportunités pour certains salariés, il est évident que cette pratique doit être encadrée pour éviter les dérives. En France, quelque 5 millions de salariés ont ainsi dû exercer leur métier à la maison du jour au lendemain, sans y être préparés et sans encadrement pour la très grande majorité d'entre elles et d'entre eux. Il est vrai que certains points doivent être réglés, mais je crois qu'inscrire dans la loi un droit pour les femmes enceintes et fixer une durée serait un véritable

Ainsi, lorsqu'ils ont moins de trois ans, seuls 41 % des enfants de foyers monoparentaux ont une mère occupant un emploi, contre 63 % des enfants vivant avec des parents en couple. Par ailleurs, les mères des foyers monoparentaux sont également celles qui supportent le plus de temps partiel subi : 47 % de celles qui ont un emploi à temps partiel souhaiteraient travailler davantage. Afin de favoriser le maintien ou la reprise d'une activité professionnelle des salariés à la tête d'une famille monoparentale, il faut proposer des solutions.

qu'il permet dans l'organisation d'une journée. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons l'encourager pour les personnes assumant seules la charge d'un ou plusieurs enfants en introduisant l'obligation pour les employeurs de motiver leur refus à une demande émanant d'un salarié à la tête d'une famille monoparentale.

Il est important de rappeler que, d'une manière générale, l'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à ce mode d'organisation doit motiver sa réponse. Il ne semble donc pas utile d'allonger davantage la liste des cas nécessitant un formalisme supplémentaire. L'avis de

pour une mise en oeuvre réussie du télétravail. Le cadre juridique existant en matière de télétravail est suffisamment souple et complet pour permettre une plus grande diffusion de cette pratique et répondre à l'aspiration à l'aspiration des salariés et des employeurs à repenser l'organisation de leur travail. Il n'est donc pas, à notre avis, opportun de modifier la loi au risque de perdre en lisibilité. Par ailleurs, il faut veiller à ne pas créer des injonctions contradictoires

inégalité, les crèches à vocation d'insertion professionnelle sont une solution efficace : elles permettent l'accueil des jeunes enfants de 0 à 3 ans de parents sans emploi, et l'accompagnement de ces derniers vers l'emploi ou la formation professionnelle. Reconnaître dans la loi l'existence de ces crèches

Cette précision nous apparaît pertinente. C'est pourquoi nous défendons aujourd'hui le rétablissement de cette disposition, afin non seulement d'encourager la création de ces crèches, mais également de nous assurer qu'elles pourront être un levier vers une meilleure accessibilité à l'emploi des parents qui en sont éloignés, en priorité des femmes. En ce sens, il apparaît que ce dispositif a toute sa place dans le texte que nous examinons.

une répartition inégale des tâches domestiques et familiales. Je rappelle que, dans une étude portant sur le temps domestique et parental des hommes et des femmes, l'Insee a établi que les femmes consacrent chaque jour 4 heures 38 aux tâches domestiques et familiales,

Par conséquent, cet amendement vise à rétablir l'article prévoyant de sensibiliser les parents à la lutte contre les stéréotypes de genre, en y ajoutant la lutte contre les inégalités de répartition des travaux domestiques et familiaux. L'Union nationale des associations familiales serait défavorable à une telle mesure

à la recherche d'une meilleure égalité entre les femmes et les hommes, objectif dont le corollaire est la lutte contre les stéréotypes de genre et l'attention portée à la question de la répartition des charges domestiques. Par conséquent, j'émettrai un avis de sagesse sur cet amendement.

prévoyaient que les formations à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques dispensées dans les écoles et les formations dispensées aux élèves dans les collèges, notamment concernant l'orientation et la découverte des métiers, contribuent à lutter contre les stéréotypes de genre. En effet, la lutte contre ces stéréotypes doit être engagée dès le plus jeune âge. Agir le plus en amont possible des choix d'orientation, en luttant contre les déterminants de genre dans l'apprentissage des compétences comme dans l'orientation professionnelle, est une condition pour atteindre la parité dans certains corps de métiers. De plus, inscrire la lutte contre les stéréotypes de genre dans l'usage des outils et des ressources numériques, mais aussi dans l'orientation professionnelle vers les secteurs de l'informatique et des nouvelles technologies, devrait contribuer à permettre aux jeunes femmes de leur ouvrir la d'aller vers ces métiers et, plus largement, d'acquérir des compétences indispensables sur un marché du travail en mutation rapide. Je rappelle que les métiers d'avenir, ceux que

de le citer, car il est très explicite : les établissements scolaires et de l'enseignement supérieur « contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation » et « assurent une mission d'information sur les violences, y compris en ligne, et une éducation à la sexualité ».

préciser l'article auquel je faisais référence. L'article L. 331-7 du code de l'éducation dispose que chaque élève bénéficie, à toutes les étapes de sa scolarité, d'« un parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel », lequel est réalisé dans le cadre d'un

M. Thierry Cozic. L'article 5 pose les bases légales préalables à la construction d'un index de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements du supérieur. Le présent amendement vise à doubler l'effort de publication d'indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes d'une obligation de transparence sur les actions menées en cas de résultats insatisfaisants, afin d'assurer la progression de l'établissement. Il est inspiré de l'expérience acquise la mise en oeuvre de l'index de l'égalité professionnelle en entreprise,

ou, lorsque le nombre de membres du jury est impair - il faut bien tout prévoir ! -, à ce que l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas

de 40 % dans les jurys et comités de sélection de la fonction publique, nous proposons de supprimer les dérogations accordées aux établissements publics de l'enseignement supérieur agricole

casser les stéréotypes selon lesquels les écoles militaires seraient exclusivement masculines, et les écoles sanitaires et sociales exclusivement féminines.

la loi ne rend pas obligatoire la mise en oeuvre de corrections. Or l'index n'a de sens que s'il entraîne par la suite une correction des inégalités de la part des employeurs. Il vaut mieux qu'une entreprise agisse en corrigeant les inégalités salariales, plutôt qu'elle maintienne les inégalités entre les femmes et les hommes en s'acquittant d'une pénalité financière.

est à Mme Guylène Pantel. L'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires impose aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 40 000 habitants une obligation de nominations équilibrées dans les emplois de direction. Dans un avis sur la parité dans les intercommunalités rendu en 2018, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes rappelait que le développement des compétences stratégiques des intercommunalités et l'accroissement de leur périmètre ont eu pour conséquence la multiplication des emplois de direction en leur sein. Toutefois la population moyenne des EPCI étant de 52 000 habitants, un grand nombre des emplois de direction des intercommunalités ne sont pas concernés par les dispositifs paritaires. cette raison, le Haut Conseil recommande que la loi Sauvadet s'applique à tous les emplois de direction des intercommunalités, sans qu'un seuil d'habitants soit imposé. Sans supprimer immédiatement le seuil de 40 000 habitants, nous proposons d'étendre l'obligation de nominations équilibrées dans les emplois de direction prévue par la loi Sauvadet

La question de l'abaissement du seuil des nominations équilibrées dans la fonction publique territoriale a été très largement discutée lors de l'examen de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, qui a déjà prévu un abaissement du seuil de 80 000 à 40 000 habitants.

coûte 90 000 euros à l'administration concernée. En 2017, Bercy a ainsi dû payer 1,7 million d'euros et, en 2020, six ministères ont été sanctionnés. Les effectifs du ministère de l'économie, des finances et de la relance sont composés à 56 % de femmes, mais seulement 30 % des postes d'encadrement sont occupés par des femmes.

donc de remplacer le taux de 40 % prévu par celui de 50 % pour les nominations prononcées après l'année 2023. La loi Sauvadet fixe des quotas en vue d'assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les nominations aux plus hauts postes de l'administration des trois fonctions publiques. Cette perspective de féminisation doit se poursuivre, jusqu'à ce que la parité soit atteinte pour répondre à l'équilibre des primo-nominations.

la commission n'est pas favorable à l'augmentation de ces quotas.

objectif a été avancé à l'année 2017. L'augmentation progressive de cet objectif chiffré a permis un bon ancrage de cette mesure. Les plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle élaborés par chaque employeur public comportent des actions visant à favoriser la création de viviers de femmes. Pour agir rapidement et concrètement en ce sens, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin, a lancé un programme de baptisé « Talentueuses ».

est à Mme Guylène Pantel. L'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires impose notamment aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan d'action pluriannuel visant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les auteurs de cet amendement proposent d'abaisser ce seuil aux collectivités territoriales et EPCI de plus de 10 000 habitants, lesquels disposent de directeurs généraux des services et de structures adéquates pour mettre en oeuvre un tel plan d'action. Il nous semble en effet essentiel que de petites collectivités territoriales, dans lesquelles les inégalités de parcours et de rémunération

qui traduisait le choix de faire porter cette obligation nouvelle par les collectivités les plus à même d'en supporter la charge organisationnelle. De la même manière que pour les amendements précédents, la commission des affaires sociales n'a pu, au cours de ses travaux, apprécier l'opportunité de modifier ces obligations dans le champ de la fonction publique ni en évaluer les effets

d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, élaborés selon des modalités et des méthodologies définies par décret. Ce dispositif permettra d'objectiver et de mesurer annuellement les résultats obtenus par les administrations publiques en matière d'égalité

à la mise en place d'indicateurs issus du RSU, afin d'objectiver et de mesurer annuellement les résultats obtenus par les administrations publiques en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces dispositions répondent également à une demande très forte des organisations syndicales et des associations des femmes de la fonction publique pour davantage de transparence sur l'égalité professionnelle dans le secteur public, à l'instar de ce que prévoit l'index pour le secteur privé. Il s'agit d'un point de départ et d'objectivation essentiel pour accélérer réellement l'égalité professionnelle et économique dans la fonction publique, qui constitue l'une des priorités de la ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin. Bien que l'article 9 9 A du statut général de la fonction publique précise le contenu du RSU, l'élaboration d'un véritable baromètre de l'égalité professionnelle,

madame la ministre,

lauréate de la 24 édition du Parlement des enfants, visant à renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, rédigée par la classe de l'école de Canto Perdrix 2 de Martigues. Cet amendement vise à insérer dans le code du sport un nouvel article posant le principe de l'égalité de rémunération des sportives et des sportifs, et des sportifs, les fédérations délégataires étant chargées d'édicter des règlements destinés à en garantir le respect par les associations et sociétés sportives placées sous leur autorité. Ce principe d'égalité des rémunérations s'applique également aux prix en argent ou en nature

le droit du travail leur est applicable, en particulier le principe de non-discrimination et celui d'une rémunération égale pour des travaux égaux. Je ne mesure pas parfaitement l'intérêt de créer un droit spécifique pour les sportifs.

et des sportifs, les clubs employeurs et les fédérations sportives sont déjà soumis aux conditions du code du travail imposant à tout employeur d'assurer, pour un même travail, de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Ce principe interdit bien évidemment toute discrimination de salaire fondée sur le sexe. En outre, dans les clubs et fédérations d'au moins cinquante salariés, l'employeur doit également publier chaque année l'index de l'égalité femmes-hommes. Enfin, les conditions de rémunération et de statut relèvent de la négociation collective entre les partenaires sociaux de la branche- convention nationale du sport, accords collectifs par discipline, voire même accords d'entreprise -et non des règlements des fédérations.

qui agissent en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mon collègue député Pierre Dharréville avait d'ailleurs déposé, le 3 novembre 2020, cette proposition de loi rédigée par la classe de Canto Perdrix 2 de Martigues. Le sport est aussi marqué par une lente évolution des mentalités de la société.

pour faire avancer l'égalité et les droits des femmes. En 2017, l'Insee a publié une enquête sur les pratiques physiques et sportives, qui révélait les inégalités persistantes entre femmes et hommes en termes de temps consacré au sport que de disciplines pratiquées. L'activité sportive révèle des inégalités de genre, notamment chez les jeunes : seulement 33 % des femmes de 16 à 24 ans pratiquent un sport une fois par semaine, soit

Beaucoup de femmes de mon âge se demandent pourquoi nous en sommes encore là. À ce rythme, si rien n'est fait, il faudra deux siècles pour parvenir à l'égalité dans la répartition des tâches ménagères.

Il est pourtant évident que les inégalités professionnelles et économiques trouvent en partie leur fondement dans l'inégale répartition des tâches domestiques. De même, si nous voulons réellement offrir des perspectives de carrière et d'indépendance économique égales selon les genres, il est tout aussi évident que nous devons sensibiliser les parents à la question de ces stéréotypes, qui sont au coeur des inégalités.

... Quel est l'avis de la commission ? L'article 5 prévoit que la formation des conseillers d'orientation devra comprendre des contenus relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les stéréotypes de genre,

À la rentrée scolaire de 2017, Jean-Michel Blanquer a créé un corps unique de psychologues de l'éducation nationale. L'annexe de l'arrêté du 26 avril 2017 définit très précisément la liste des connaissances et des compétences professionnelles que les psychologues de l'éducation nationale doivent avoir pour exercer leur métier. Je veux vous rassurer, madame la sénatrice : ce référentiel de connaissances et de compétences prévoit déjà un objectif de réussite de tous les élèves dans une indispensable complémentarité de la mission d'enseignement et de l'action éducative de l'école. éducative de l'école. Les élèves et les étudiants peuvent également bénéficier d'un accompagnement spécifique dans l'élaboration de leur projet d'avenir et d'un conseil en orientation, notamment en créant les conditions qui favorisent leur capacité à se distancier des stéréotypes professionnels, qu'ils soient sociaux ou de genre. La formation initiale des psychologues de l'éducation nationale s'appuie sur ce référentiel de connaissances et de compétences. Elle comprend aussi une unité d'enseignement sur les thèmes du genre, de la scolarité, de l'orientation et du travail, dont les objectifs sont de développer la capacité d'analyse des causes et des effets de la division sexuée et de l'orientation du travail, d'être en mesure de questionner le rôle de l'école, des politiques, des procédures et des pratiques de l'éducation à l'orientation. Il s'agit aussi de développer la réflexion sur le rôle de psychologue de l'éducation nationale et sur les pratiques qui peuvent être mises en oeuvre pour contribuer à la « désexuation

devraient se saisir afin de prendre en compte et de lutter contre les biais de genre, en raison desquels certaines élèves ne se sentent pas légitimes à intégrer certaines formations. La

Nous nous félicitons que ces critères soient déjà pris en considération dans les règlements internes et nous pourrions même nous en satisfaire si les inégalités entre les femmes et les hommes dans les écoles d'ingénieurs ne demeuraient pas aussi fortes. Je rappelle qu'en 2019, selon les chiffres du ministère de l'enseignement supérieur, seulement 28 % des élèves inscrits dans les formations d'ingénieurs étaient des femmes. Eu égard aux résistances des formations scientifiques, notamment

parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, un cinquième indicateur existe : l'écart du taux de promotion entre les femmes et les hommes. Cet index est un outil précieux, car il permet de mettre en lumière des dysfonctionnements et de constater que nous sommes encore loin de l'égalité salariale. Du chemin reste à faire ! La parole

Depuis le début du quinquennat, nous avons mis en oeuvre des mesures fortes pour résorber cet écart inacceptable. L'index de l'égalité professionnelle, mis en place par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est un outil puissant pour faire changer durablement les pratiques, parce qu'il impose une obligation de résultat et un référentiel commun permettant de noter et de classer les entreprises. Les résultats des premiers exercices montrent que l'index modifie les comportements, année après année. En 2021, la note globale continue de progresser, passant de 84 à 85. 85. Mieux, la note moyenne des entreprises de plus de 1 000 salariés est passée de presque 83 en 2019 à plus de 88 en 2021, ce qui représente une réelle progression.

D'une part, l'inscription dans la loi de l'obligation de publier l'ensemble des indicateurs qui composent l'index permettra d'inciter les entreprises à renforcer leurs actions en matière d'égalité femmes-hommes. Je crois que la transparence est un outil puissant pour faire changer les pratiques. l'article 6 prévoit également que les entreprises devront désormais se fixer et publier des objectifs de progression pour chaque indicateur, dès lors que la note obtenue à l'index sera en deçà d'un certain seuil. Cette disposition doit encourager les entreprises à engager concrètement le changement et à modifier leur politique de rémunération en profondeur. Par ailleurs, les entreprises qui sont le plus en retard- celles qui ont encore un index inférieur à 75 points -devront désormais publier les mesures de correction adoptées. Là encore, cela doit renforcer la transparence sur les efforts mis en oeuvre par les entreprises afin d'améliorer les pratiques. Ainsi, avec cet article, les entreprises qui ont encore des marges importantes de progrès en matière d'égalité salariale devront se doter d'objectifs clairs, chiffrés et concrets. Tout en veillant à ne pas introduire trop de complexité pour nos entreprises, nous souhaitons au travers de cet article tracer dans chaque structure un horizon clair pour une meilleure égalité, connu non seulement de tous les salariés mais également des partenaires extérieurs de l'entreprise. C'est là l'égalité des chances en acte : veiller à ce que les objectifs fixés collectivement

les limites actuelles de l'index de l'égalité femmes-hommes, institué en septembre 2018, et suggère d'en améliorer l'efficacité. Parmi les carences relevées, il est précisé que l'index ne tient pas compte des différences de temps de travail. Or ne pas recenser les temps partiels revient à effacer des différences structurelles essentielles, puisque, on le sait, le temps de travail compte pour beaucoup dans la fabrique des inégalités de rémunération entre hommes et femmes. En effet, 85 % des salariés à temps partiel sont des femmes. Ainsi, au travers de cet amendement, nous souhaitons compléter cet index afin qu'il tienne compte non seulement des écarts de rémunération mais également des différences de temps de travail.

Madame la sénatrice, le Gouvernement partage votre volonté de prêter une attention particulière aux salariés à temps partiel, parmi lesquels les femmes sont surreprésentées puisqu'elles occupent quatre emplois à temps partiel sur effectivement être utile de mieux mettre en lumière la part des femmes parmi les salariés en contrats courts ou à temps partiel dans les entreprises. Pour autant, cette donnée n'a pas vocation à relever de l'index, lequel, pour plus de lisibilité, se concentre sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Pour cette raison, le Gouvernement est également défavorable à l'amendement.

Nous pensons que l'index peut être un outil pour montrer l'exemplarité de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière, l'objectif étant de démontrer l'absence d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. un devoir d'exemplarité de la République, laquelle ne saurait admettre quelque exception que ce soit. Le suivi des dispositifs paritaires aujourd'hui mis en place est souvent insuffisant et ne permet pas de s'assurer que les mesures sont effectivement mises en oeuvre. La connaissance la plus large possible des avancées en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est une première étape vers la réalisation d'une égalité effective.

Cette proposition est satisfaite puisque le ministère du travail- je parle sous votre contrôle, madame la ministre -collecte déjà les résultats des entreprises, notamment le réseau déconcentré des inspections du travail

aux mesures liées au code de commerce, elles sont suivies par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, notamment par la direction générale du Trésor, la direction générale des entreprises et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression

les entreprises qui n'auraient pas réussi à corriger leurs insuffisances se verraient en effet frappées d'une pénalité, n'est pas encore échu. Quoique je partage votre ambition, Mme Cohen, sur le principe, on ne peut pas faire comme si les entreprises n'avaient pas traversé une période

En effet, la négociation des accords salariaux au sein des entreprises et la publication des écarts de rémunération constituent une première étape ; la deuxième étape consiste à rendre obligatoire telle négociation dans les entreprises, ainsi que la mise en oeuvre d'un plan pour l'égalité professionnelle dans les entreprises où des écarts sont constatés. Il s'agit de passer d'une obligation de moyen à une obligation de résultat.

de loi, nous proposons de passer d'une simple incitation à une obligation en matière de plan pour l'égalité professionnelle au sein des entreprises, comme vient de le souligner ma collègue Cathy Apourceau-Poly.

prévoit aujourd'hui que l'employeur peut prendre des mesures visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans un deuxième temps, ces mesures peuvent faire l'objet d'une négociation au sein de l'entreprise en vue de l'élaboration d'un plan d'action pour l'égalité professionnelle.

En réalité, les quotas de femmes dans les comités exécutifs, c'est bien ; mais, pour les filles qui sont à l'usine ou pour les femmes qui travaillent comme

à l'Assemblée nationale se préoccupent de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ! L'index de l'égalité professionnelle est une réelle avancée, dont on peut mesurer année après année l'effet sur le changement des comportements.

un rattrapage égal à la moyenne des augmentations accordées aux salariés de même qualification. Mais ces obligations ne sont pas toujours respectées, loin de là. Selon le ministère du travail, 29 % des entreprises ne les respectent pas. Si des sanctions Si des sanctions sont prévues- l'entreprise risque une amende de 1 500 euros, doublée en cas de récidive -, il semblerait, au vu des chiffres, que celles-ci ne soient pas suffisamment dissuasives. Nous proposons donc de renforcer les sanctions applicables à ceux qui n'appliquent pas la loi.

à davantage de postes à responsabilité. Alors que la loi Copé-Zimmermann visait les conseils d'administration et de surveillance, qui déterminent les orientations générales de l'activité de la société, nous visons, avec cette proposition de loi, les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, c'est-à-dire celles et ceux qui prennent au jour le jour les décisions opérationnelles opérationnelles et assurent la direction effective de l'entreprise. En outre, alors que les membres des conseils d'administration et de surveillance sont généralement recrutés en externe, il s'agit désormais aussi de faciliter, pour les femmes, l'accession

des quotas. La loi Copé-Zimmermann a prouvé non seulement que les quotas fonctionnaient, mais aussi que le vivier de femmes compétentes pour intégrer de tels postes existait. Cette féminisation ne s'est pas seulement révélée bénéfique pour la gouvernance ; elle l'a été également pour la performance économique des entreprises.

est à Mme la ministre. L'article 7 doit nous permettre de changer la donne en faveur d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les titulaires des postes à plus haute responsabilité des entreprises. La situation actuelle est en effet loin d'être satisfaisante. Les femmes ne représentent aujourd'hui que 18 % des membres des comités exécutifs des entreprises du CAC 40, alors même qu'elles représentent un tiers des cadres. Une seule femme est directrice générale d'une entreprise du CAC 40. J'ajoute que les résultats de l'indicateur de l'index relatif à la parité parmi les dix plus hautes rémunérations témoignent d'une dégradation : 37 % des entreprises de plus de 1 000 salariés moins de deux femmes parmi les dix plus hautes rémunérations en 2020 ; elles sont 43 % cette année ! Il est donc nécessaire de prendre des mesures fortes pour faire évoluer durablement les pratiques. C'est toute l'ambition de cet article 7 qui, je le crois, va donner une impulsion décisive en faveur de la parité entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Il prévoit, d'une part, une nouvelle obligation de publication relative aux écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes

ans. Visant à la fois les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, cet article permet un renouvellement en profondeur et dans la durée des viviers d'hommes et de femmes qui occupent aujourd'hui et occuperont demain les postes à haute responsabilité dans l'entreprise. Il faut bien le dire, il s'agissait là d'un angle mort de nos politiques d'égalité au sein de l'entreprise. La loi Copé-Zimmermann a fait beaucoup concernant la parité dans les conseils d'administration et de surveillance et personne aujourd'hui ne la remet en cause ; il était donc temps d'avancer pour les postes de direction opérationnelle dans les entreprises.